La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 septembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 1 septembre 2021 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 20 septembre 2021. Acte est donné de cette communication. Ce décret a été publié sur le site internet du Sénat. En conséquence, je constate que la troisième session extraordinaire de 2020-2021 est ouverte. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c'est avec émotion que nous avons appris le décès, jeudi 9 septembre dernier, de notre ancienne collègue Lucette Michaux-Chevry, vaincue par la maladie contre laquelle elle luttait avec le courage et la détermination qui la caractérisaient. Figure majeure de la vie politique guadeloupéenne depuis 1959, date de sa première élection comme conseiller municipal de Saint-Claude, elle assumera ensuite tous les mandats qui ponctuent le d'un élu de terrain. Élue conseillère générale en 1976, elle devient présidente de l'assemblée départementale en 1982. En 1987, elle se présente aux élections municipales dans la commune de Gourbeyre, dont elle devient maire. Elle le restera jusqu'en 1995. À cette date, elle part à la conquête de la ville de Basse-Terre, chef-lieu de la Guadeloupe. Elle l'emporte et en devient le premier magistrat. Elle le restera jusqu'en 2001, puis le redeviendra de 2008 à 2014. En 1992, elle remporte l'élection régionale et prend en main les destinées du conseil régional. Elle conservera ce poste jusqu'en 2004. C'est dire la place importante qu'occupait notre ancienne collègue auprès de ses concitoyens. étant, son rayonnement dépassait largement les limites de l'archipel guadeloupéen. Elle poursuit son engagement politique à l'Assemblée nationale, où elle est élue députée en 1986, puis de 1988 à 1993. En 1995, elle entre au Sénat. Elle siégera dans cet hémicycle jusqu'en 2011. Ceux qui l'ont côtoyée se souviennent de sa maîtrise de l'art oratoire, de sa force de persuasion et de ses convictions fortes. Ils se souviennent notamment de son intervention lors de l'hommage solennel à Victor Schoelcher. À cette occasion, elle rappela que la France ne pouvait se contenter d'un devoir de mémoire, mais se devait de donner à son espace géographique historique sa vraie dimension, sans persister dans une vision restrictive, limitée à l'Hexagone. Pour elle, la France, c'était beaucoup plus ! Parallèlement, Lucette Michaux-Chevry défend, bien avant que celle-ci ne devienne un sujet d'actualité, la différenciation territoriale comme levier de développement des outre-mer. La déclaration de Basse-Terre, qu'elle cosigna avec les présidents d'exécutifs de Martinique et de Guyane, a jeté les bases de cette politique. Ce parcours exceptionnel d'une femme engagée n'aurait pas été complet si elle n'avait exercé par deux fois des fonctions ministérielles de 1986 à 1988 comme secrétaire d'État à la francophonie, puis de 1993 à 1995 comme ministre déléguée chargée de l'action humanitaire et des droits de l'homme. Au nom du président du Sénat et du Sénat tout entier, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille et à ses proches. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, présentée par Mme Nathalie Goulet (proposition n° 674, texte

Cette réforme doit entrer en vigueur à compter des élections de 2022. Or, dans le même temps, le législateur a modifié par mégarde les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge consulaire. le rappelle, ces dernières étaient, jusqu'à présent, calquées sur les conditions imposées pour participer à l'élection des délégués consulaires. L'une des conséquences de cette modification est que les juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes ne sont plus rééligibles en cette seule qualité. Il en va de même des anciens membres de ces tribunaux. Autrement dit, si elle était mise en oeuvre en l'état, cette modification des conditions d'éligibilité aurait des conséquences fort dommageables pour les tribunaux de commerce. Songez en effet qu'elle priverait les tribunaux d'un vivier de candidats assez considérable. Pour la seule année 2021, de 450 à 500 des 793 juges consulaires dont le mandat arrive à expiration deviendraient inéligibles si la loi n'était pas modifiée. serait d'autant plus préjudiciable qu'il s'agit, en général, des magistrats les plus confirmés et les plus expérimentés, parmi lesquels- naturellement -le président du tribunal est très souvent choisi. s'agit donc d'une évidence : les tribunaux de commerce ne peuvent tout simplement pas se passer de leurs services. C'est ce qui a conduit notre collègue Nathalie Goulet à déposer cette proposition de loi, laquelle vise à rétablir l'éligibilité des juges consulaires en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes. Notre commission des lois a adopté ce texte à l'unanimité, en y apportant toutefois quelques modifications et quelques compléments. Tout d'abord, il nous a paru opportun de rétablir l'éligibilité des anciens juges. Précédemment, une cinquantaine de membres des tribunaux de commerce, aujourd'hui en fonctions, s'étaient portés candidats en tant qu'anciens juges, en tout cas selon les informations dont nous disposons. Il serait également dommageable de se priver de telles compétences. De plus, notre commission a rétabli les inéligibilités liées à certaines condamnations pénales et civiles, qui, elles aussi, se sont malencontreusement perdues en chemin lors de l'examen de la loi Pacte.

plafonnement a été privé d'effet par une interprétation, du reste contestable, du Conseil d'État. En outre, la commission a précisé les dispositions relatives au corps électoral des juges consulaires. Il s'agissait principalement d'élever au rang législatif des dispositions introduites par décret et, pour cette raison, juridiquement fragiles, même si elles paraissaient opportunes sur le fond. De même que les conditions d'éligibilité, les conditions de participation à l'élection des juges des tribunaux de commerce relèvent, en effet, du domaine de la loi, en tant que règles constitutives d'un ordre de juridiction, en application de l'article 34 de notre Constitution. S'agissant du calendrier électoral, la commission a prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016, afin de tenir compte du report de plusieurs semaines des élections des juges consulaires cette année.

je suis très heureux d'être de retour parmi vous au Sénat, après la trêve estivale, pour débattre d'un sujet crucial pour notre économie je veux bien sûr parler de la justice commerciale. Ce que l'on appelle aussi « justice consulaire » est une institution du système judiciaire français vieille de plus de cinq siècles. Une telle

Plus que jamais au cours de ces derniers mois de crise sanitaire, les tribunaux de commerce ont répondu présent dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Le « quoi qu'il en coûte » décidé par le Président de la République a permis de préserver de manière exceptionnelle notre économie au pire de la crise sanitaire.

pendant la crise sanitaire laisseront place au fonctionnement normal et ordinaire de l'économie. Je pense par exemple à la toute nouvelle procédure de traitement de sortie de crise, qui va entrer en vigueur au début du mois d'octobre prochain. Cette procédure novatrice permettra, j'en suis sûr, d'éviter un grand nombre de faillites, en intervenant le plus tôt possible auprès de l'entreprise en difficulté. Le succès de ces nouvelles dispositions reposera largement sur les juridictions commerciales. C'est pourquoi le Gouvernement est particulièrement soucieux de donner aux tribunaux de commerce les moyens de remplir leurs missions avec efficacité et diligence. L'une des spécificités de la justice commerciale est qu'elle repose sur le bénévolat de ses juges. C'est une justice de proximité, peut-être même la justice de proximité par excellence et par définition. En effet, elle est à la fois proche géographiquement et sociologiquement de ses justiciables, car ses juges viennent directement du tissu économique local. C'est pour ces raisons, couplées au besoin vital de disposer d'une justice consulaire pleinement opérationnelle, que, sans faire durer un suspense insoutenable, le Gouvernement apporte son soutien

En effet, elle permet de conserver les juges les plus expérimentés, les plus capés, au sein de nos juridictions, alors que la justice commerciale sera probablement très sollicitée dans les mois à venir. continuer à bénéficier des compétences reconnues de ces juges et de leurs connaissances, acquises au cours de leurs précédents mandats. Soyons précis. Nos tribunaux de commerce comptent actuellement 3 357 juges consulaires. Or 793 d'entre eux voient leur mandat se renouveler cette année, soit 23 % des effectifs, répartis en 134 tribunaux de commerce et 31 cours d'appel. Tous les tribunaux de commerce et tribunaux mixtes de commerce sont concernés, des tribunaux de commerce d'Alençon et d'Arras à ceux de Villefranche et Saint-Pierre de La Réunion. Parmi les plus importants en nombre de juges consulaires, on peut citer Paris, Nanterre, Aix-en-Provence, Évry ou encore Créteil. Parce que la fonction de juge de commerce demande une implication forte et un engagement particulièrement chronophage, nombre de ces juges sont retraités ou décident de se consacrer pleinement à leurs fonctions. Or, en l'état actuel du droit, près de 472 juges consulaires, soit environ 14 % des effectifs, ne pourraient être candidats aux prochaines élections du fait des nouvelles conditions d'éligibilité. Une telle perte de compétence, d'expérience et de savoir-faire serait d'autant plus regrettable que ces juges expérimentés occupent la plupart du temps des fonctions importantes, comme celles de président ou de président de chambre. Elle serait aussi dommageable, parce que la qualité reconnue des juges consulaires est un véritable atout et un facteur d'efficacité de nos juridictions commerciales. Ces juges doivent donc pouvoir se présenter aux prochaines élections consulaires : c'est pourquoi il est nécessaire que le Parlement adopte le présent texte suffisamment en amont des élections qui auront lieu prochainement. Pour nous permettre à tous d'avancer avec vitesse, mais sans précipitation, j'ai repoussé par décret la date des élections consulaires, qui se dérouleront entre les 22 novembre et 5 décembre

par votre rapporteur et votre commission des lois, qui ont enrichi encore la proposition de loi par des mesures nécessaires et consensuelles, défendues par le Conseil national des tribunaux de commerce comme par la conférence générale des juges consulaires de France, et soutenues par la Chancellerie, en vue

: s'assurer que les juges consulaires sortants, ainsi que, sous certaines conditions, les anciens juges des tribunaux de commerce puissent se présenter aux prochaines élections.

dans les périodes difficiles. Ils méritent l'entier soutien du Gouvernement en faveur de cette proposition de loi.

de simplification, une loi de modernisation de la justice soutenue par la Haute Assemblée a étendu la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans, reconnaissant ainsi le rôle de cette institution spécialisée. Cette reconnaissance s'accompagnait bien sûr d'une possibilité nouvelle pour les mêmes artisans d'être électeurs et élus au sein de ces juridictions. M. le rapporteur l'a rappelé : peu de temps après, la loi Pacte, se voulant simplificatrice, a réformé les modalités de des juges consulaires, désormais élus par les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, en plus des juges et anciens juges du tribunal. Toutefois, en recomposant le corps éligible pour exercer les fonctions de juge, on a omis les juges et anciens juges du tribunal et des tribunaux limitrophes.

s'inscrit dans la lignée du récent rapport dédié aux outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l'aune de la crise de la covid-19, préconisant de renforcer le rôle et la spécialisation

2 du présent texte, lequel permet d'éviter une trop grande professionnalisation en limitant à cinq mandats la possibilité, pour un juge, d'exercer dans un même tribunal. Ainsi, on a bien fait le choix de privilégier des juges toujours impliqués dans le monde de l'entreprise.

Nous resterons attentifs à l'équilibre obtenu en commission. Oui, il était capital d'assurer le corps électoral et éligible le plus représentatif du monde de l'entreprise. Il était tout aussi important

Vous le savez : depuis le décret d'août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, ces juridictions de premier degré sont composées de juges consulaires élus par un collège électoral lui-même composé des délégués consulaires élus, des juges du tribunal déjà en poste et des anciens membres du tribunal inscrits sur la liste électorale. Les juges consulaires représentent aujourd'hui plus de 3 300 femmes et hommes issus du monde de l'entreprise- chefs d'entreprise, dirigeants ou cadres supérieurs -élus par leurs pairs, qui se mettent bénévolement au service de la justice commerciale. Répartis dans 134 tribunaux de commerce, auxquels s'ajoutent les tribunaux mixtes d'Alsace-Moselle et d'outre-mer, ces juges consulaires sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales, aux actes de commerce entre toutes personnes, aux billets à ordre, et sur les procédures de mandat, de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et de rétablissement personnel. Garants de la justice commerciale, ces juges doivent décider du sort de milliers d'entreprises en difficulté ainsi que du destin de centaines de milliers d'emplois. Pour exercer ces fonctions, ils tirent toute légitimité de leur élection par leurs pairs et par les représentants du monde économique. Récemment encore, l'élection des juges consulaires, encadrée par le code de commerce, reposait sur un scrutin à deux tours. Les juges étaient désignés par un collège électoral composé pour l'essentiel des délégués consulaires, des délégués consulaires, élus eux-mêmes pour une durée de cinq ans par les entrepreneurs individuels ayant le statut de commerçant ou d'artisan, les représentants des sociétés commerciales ayant leur siège ou un établissement dans le ressort du tribunal, ainsi que les cadres dirigeants employés par ces entrepreneurs ou ces sociétés, principalement. Le collège électoral comprenait également les juges du tribunal de commerce de la circonscription, ainsi que d'anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 40 de la loi Pacte a remplacé ce scrutin indirect par une élection directe par les membres élus des CCI et des CMA dans le ressort de la juridiction, ainsi que par les juges et anciens juges du tribunal de commerce. Cette disposition entrera en vigueur à la fin du mandat des délégués consulaires élus en 2016. Toutefois, ces nouvelles modalités écartent de l'éligibilité les membres en exercice et les anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes.

Une autre erreur de la loi Pacte a été corrigée par le rétablissement de l'inéligibilité des personnes condamnées pénalement. Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, la commission a introduit d'autres dispositions précisant l'électorat et l'éligibilité des juges consulaires. À titre d'exemple, l'article 2 limite à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu'une même personne peut assumer en tant que juge consulaire dans un même tribunal.

L'article 3 apporte plusieurs précisions aux conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires. Enfin, l'article 4 tire les conséquences, d'une part, du report

nous semblent également aller dans le bon sens. L'un d'eux tend à permettre aux préfectures de solliciter le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats aux élections des juges consulaires, afin de vérifier s'ils sont effectivement éligibles.

chers collègues, l'immense travail de modernisation de la juridiction commerciale passera aussi par le renforcement des garanties entourant le statut des juges consulaires, ainsi que par le parachèvement de la spécialisation de certains tribunaux de commerce. À l'avenir, nous serons sûrement appelés

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun le sait ici, ce serait une erreur de voir dans ce texte à l'apparence technique une loi sans intérêt véritable. En écho aux écrits du philosophe Gilbert Simondon, les objets techniques ne doivent nullement être dévalués comme des choses de second rang : ils sont la condition du bon fonctionnement d'un système entier, en ce qu'ils permettent son accomplissement cohérent. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet contribue à assurer la cohérence de notre législation sur un point dont les enjeux ne sauraient être minorés.

Suivant les estimations indiquées, cela représenterait entre 450 et 500 juges consulaires, sur les 793 juges ne pouvant être réélus. Une telle conséquence n'avait naturellement pas été souhaitée par le législateur, d'autant que, par tradition, les juges du tribunal de commerce sont des magistrats élus par leurs pairs parmi les commerçants ou dirigeants des sociétés commerciales. Les tribunaux de commerce sont parmi les juridictions françaises les plus ancrées dans leur particularisme historique. Il est impératif de ne pas nuire au bon fonctionnement de cette institution, donc de ne pas perdre autant d'hommes et de femmes ayant déjà montré leur compétence et leur intérêt pour leur juridiction. Cette proposition de loi vise donc, en son article 1, à modifier l'article L. 723-4 du code de commerce désignant les personnes éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, en y intégrant les membres en exercice et anciens membres. Nous ne pouvons que suivre l'évolution souhaitée, puisque, actuellement, à la lecture du code, ne sont éligibles que les juges d'un tribunal de commerce qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus. Cela provoquerait les conséquences que nous disions précédemment. Une réforme est donc nécessaire. Nous saluons également le travail effectué par notre commission des lois, qui est allée au-delà du texte initial en rendant également éligibles les anciens juges, de sorte que soient éligibles les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce, dans quelque juridiction qu'ils aient exercé.

Le Conseil d'État est venu offrir une interprétation des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle, dite « loi J21 », et de la loi Pacte s'agissant de la limitation à cinq mandats pouvant être exercés par un juge dans un même tribunal. Suivant sa lecture des textes, l'inéligibilité ne s'appliquerait que si les mandats ont été continus. Or, comme l'ont rappelé les précédents orateurs, un tel dispositif demeurera inefficace au regard de l'objectif fixé d'éviter toute forme de professionnalisation de la fonction de juge consulaire. Nous rejoignons donc la position de la commission des lois limitant strictement à cinq le nombre de mandats pouvant être exercés par un juge dans un même tribunal. tribunal. Nous considérons également comme opportuns les ajustements effectués sur les conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires. Vous comprendrez, au regard de ces éléments, que notre groupe se prononcera unanimement en faveur de cette proposition de loi. La parole

excellente proposition, prévoyant de rendre les juges en exercice d'un tribunal de commerce de nouveau éligibles aux fonctions de juges consulaires. Avant l'entrée en vigueur, en octobre 2021, d'une disposition issue de la loi Pacte, les juges consulaires étaient en effet élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les délégués consulaires. Depuis cette loi, la qualité de délégué consulaire a été supprimée et l'éligibilité des juges consulaires modifiée. Sont désormais éligibles les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers de l'artisanat, ainsi que les juges des tribunaux de commerce non limitrophes. C'est donc par erreur, et de manière non intentionnelle, les juges et anciens juges du tribunal et des tribunaux limitrophes. Ainsi, selon ses dispositions, plus de 450, voire plus de 500 bénévoles expérimentés ne seraient plus éligibles, ce qui serait évidemment préjudiciable au bon fonctionnement des juridictions. Le texte proposé par notre collègue Nathalie Goulet vient corriger cette défectuosité législative. Comme à son habitude, la commission des lois, par l'entremise de notre collègue rapporteur, François Bonhomme, est venue parfaire l'oeuvre de la sénatrice Nathalie Goulet en adoptant quatre amendements qui font l'objet d'un large consensus, du côté tant des parlementaires que du Gouvernement.

Deux dangers opposés guettent l'économie française : la défaillance et la disparition de nombreuses entreprises viables et le risque de voir se multiplier les entreprises « zombies », c'est-à-dire les entreprises non rentables. L'ensemble des procédures judiciaires ou extrajudiciaires de traitement de l'insolvabilité ou du risque d'insolvabilité des entreprises jouent un rôle déterminant pour restructurer le passif des entreprises en difficulté, réorganiser leur structure productive et opérer un tri entre les entreprises viables et non viables. L'existence de juridictions spécialisées, composées de magistrats non professionnels issus du monde de l'entreprise, compte parmi nos atouts. Mais il faut mieux juger et continuer de moderniser la juridiction commerciale, en faisant tout d'abord évoluer les modalités d'élection des juges consulaires. La proposition de loi de Mme Nathalie Goulet permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce fait écho à la recommandation n° 46 du rapport d'information de nos collègues François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi de « mieux encadrer la participation des anciens juges du tribunal au corps électoral des juges consulaires il s'agit de remédier à un effet indésiré de la réforme récente du mode d'élection des juges consulaires issue de la loi Pacte, qui prévoit notamment le non-renouvellement des délégués consulaires. Auparavant, les juges consulaires étaient élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les délégués consulaires. La suppression du statut de délégué consulaire s'est notamment traduite par l'abrogation d'une disposition qui prévoyait la liste des personnes éligibles à ce statut. Dans celle-ci étaient mentionnés les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un juge en exercice, ou un ancien juge qui n'est donc plus inscrit sur les listes des chambres de commerce et d'industrie

c'est-à-dire 450 juges consulaires, donc une justice commerciale moins efficace. La proposition de loi vise à mettre fin au tarissement du vivier des juges consulaires. Elle tend vers une des effectifs, si j'ose dire. En effet, une bonne justice, c'est une justice qui ne manque pas de juge.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette troisième session extraordinaire s'ouvre avec l'examen d'un texte utile, puisque la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet vient remédier à un manquement de la loi Pacte. Elle vise à rétablir l'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes. Tels que nous les connaissons aujourd'hui, les tribunaux de commerce sont les héritiers d'une longue tradition. Déjà, au Moyen Âge, lors des grandes foires, les commerçants élisaient ceux d'entre eux qui seraient institués juges, afin de régler leurs différends. Les juridictions consulaires ont été créées par un édit de 1563 du roi Charles IX, pris sur l'initiative de son chancelier Michel de L'Hospital, dont la statue de marbre domine cette tribune. Il s'agissait alors de donner aux marchands un outil souple de règlement de leurs litiges. En 1673, Colbert généralisé les tribunaux consulaires à la France entière et, en 1721, il en existait déjà 73. La Révolution française a conservé le principe de ces juridictions, qui prirent, par la loi des 16 et 24 août 1790, le nom des tribunaux de commerce, qu'elles ont gardé. Elles sont l'une des rares institutions à avoir survécu à la Révolution et traversé tous les régimes. Alors que les juges des tribunaux de commerce étaient élus directement par les commerçants, à partir de 1961, c'est un collège composé de délégués consulaires, ainsi que des juges consulaires en exercice et des anciens juges du tribunal concerné, qui procède à leur élection. Toutefois, la loi Pacte a opéré une réforme des modalités d'élection des juges consulaires qui doit entrer en vigueur le 2 novembre prochain. des chambres de métiers et de l'artisanat, les CMA, en plus des juges et anciens juges du tribunal. Or la loi Pacte n'a pas prévu l'éligibilité des membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes. C'est pourquoi l'initiative de notre collègue apparaît bienvenue. Je me félicite que la commission ait enrichi le texte initial, en rendant éligibles les anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes, sous certaines conditions, et en rétablissant l'inéligibilité liée à certaines condamnations.

du nombre de mandats qu'un juge consulaire peut exercer dans le même tribunal, mais également des mesures d'ajustement de la composition du corps électoral des juges consulaires, ainsi que de la prorogation du mandat des délégués consulaires élus en 2016. Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue François Bonhomme. Cette proposition de loi apporte une réponse fort opportune à une imperfection de la loi Pacte en permettant d'éviter « un tarissement du vivier des juges », comme le relève à juste titre l'exposé de ses motifs.

la loi Pacte a modifié le mode de scrutin des juges consulaires. Ces derniers sont élus non plus par les juges en exercice, les anciens juges et les délégués consulaires, mais par les membres des CCI et CMA. Or, en supprimant les délégués consulaires, la loi Pacte a malheureusement, dans le même temps, supprimé les juges consulaires en exercice et les cadres dirigeants de la liste des personnes éligibles à la fonction de juge consulaire. La présente proposition de loi vise à corriger cet oubli. L'absence de ces candidats pour le prochain renouvellement des juges consulaires entraînerait l'éviction d'environ 450 à 500 d'entre eux, qui ne seraient pas rééligibles, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021, soit plus de la moitié. Si je prends l'exemple de mon département d'Indre-et-Loire pour illustrer mon propos, le tribunal de commerce de Tours compte 25 juges consulaires dont 11 sont renouvelables. Si la loi n'était pas modifiée, la moitié de ces 11 juges consulaires ne pourrait pas se représenter, dont le président lui-même, les présidents des deux chambres des procédures collectives et le président de l'une des trois chambres de contentieux. Cela confirme, s'il en était encore besoin, la difficulté décrite au niveau national, et l'urgence de la situation. Comme vous le savez, mes chers collègues, il faut en moyenne deux ans pour former un juge consulaire. Il faut réparer cet oubli pour conserver la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles essentielles. La présente proposition de loi proposait uniquement de modifier l'article L. 723-4 du code de commerce pour rétablir l'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes. Je souhaite saluer ici le travail de la commission des lois et de son rapporteur, notre collègue François Bonhomme, qui ont modifié le texte proposé, afin de rendre éligibles, sous certaines conditions, l'ensemble des membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce. La commission a également profité de ce texte pour rétablir l'inéligibilité des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ainsi que pour limiter à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu'une même personne peut exercer en tant que juge consulaire dans un même tribunal. Ces modifications vont dans le bon sens. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera ce texte essentiel pour le bon fonctionnement de nos tribunaux de commerce. La parole

C'est à ce principe simple que répond la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet, permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce que nous examinons aujourd'hui. En effet, la loi Pacte du 22 mai 2019 a abrogé le statut de délégué consulaire, prévoyant que le mandat de ceux qui le détenaient ne serait pas renouvelé une fois arrivé à échéance, en novembre 2021. Elle a donc malencontreusement privé d'éligibilité les membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes, sans que cela ait été souhaité par le législateur- les juges des tribunaux non limitrophes restant, eux, éligibles. Eh oui ! De ce fait, entre 450 et 500 juges consulaires, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021, pour un total de 3 357 juges consulaires en exercice, ne seraient pas rééligibles. Pour rappel, ces juges consulaires sont les juges statuant en première instance dans les tribunaux de commerce. Ils sont, ou ont été, chefs d'entreprise et statuent face à leurs pairs à titre bénévole, et je tiens ici à rendre hommage à leur engagement. Ainsi, la suppression du statut de délégué consulaire s'est traduite par l'abrogation de plusieurs articles du code de commerce, parmi lesquels l'article L. 713-7, qui prévoyait la liste des personnes éligibles au statut de juge consulaire. Au nombre de celles-ci étaient mentionnés « les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ». Or la nouvelle rédaction de l'article L. 723-4 ne mentionne plus la catégorie des juges consulaires en exercice. La présente proposition de loi vise donc à rétablir l'éligibilité des juges consulaires actuellement en poste. Car sans ce texte, environ 60 % des juges en exercice parmi les plus expérimentés ne seraient plus éligibles. sans aucun doute extrêmement dommageable pour le fonctionnement des juridictions de devoir se passer des services de ces magistrats expérimentés. En outre, sur l'initiative du rapporteur, que je salue et dont je salue le travail, la commission des lois a profité de l'examen de cette proposition de loi pour apporter diverses autres améliorations au régime électoral des juges consulaires : Elle a rétabli l'inéligibilité des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, frappées d'une peine complémentaire d'interdiction professionnelle ou sanctionnées civilement au titre de législations étrangères relatives à l'insolvabilité des entreprises, équivalentes à la législation française. Elle a ensuite limité à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu'une même personne peut exercer

en imposant notamment aux anciens juges, pour être électeurs, d'avoir exercé leurs fonctions pendant au moins six années, de n'avoir pas été déclarés démissionnaires et de ne pas être frappés d'inéligibilité. Ce texte s'inscrit pleinement dans les réflexions de la mission d'information sénatoriale sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l'aune de la crise de la covid-19, qui préconisait, à raison, de renforcer les garanties entourant le statut des juges consulaires. la proposition de loi entend remédier au problème du tarissement du vivier des juges consulaires induit par l'évolution législative de 2019. D'ailleurs, comme l'ont justement souligné le rapporteur

entreprises est primordial. L'objectif de cette proposition de loi est de corriger une malfaçon de la loi Pacte du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

des anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes. Par ailleurs, la commission a apporté diverses améliorations au régime électoral des juges consulaires, aux articles 1, L'article 4 de la proposition de loi, introduit par la commission sur l'initiative du rapporteur, vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016. Cela permettra aux élections prévues en novembre et décembre 2021 de se tenir selon les anciennes règles.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique (texte de la commission, n° 733, rapport n° 732) et des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010

le texte que nous examinons aujourd'hui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le 1 juillet dernier. Il comprend certaines avancées sur lesquelles je reviendrai, mais, il faut le rappeler, il demeure très éloigné des attentes que nous nourrissions, les uns et les autres, au début du quinquennat. Disons-le clairement, ce projet de loi n'est pas celui qui permettra au secteur de l'audiovisuel de s'adapter au monde nouveau forgé par les plateformes. Au déséquilibre des moyens s'ajoute une iniquité concernant les réglementations applicables, qui contraint le développement international des médias français. La réforme de l'audiovisuel public restera, par ailleurs, l'occasion manquée de ce quinquennat, de même que la modernisation de la contribution à l'audiovisuel public, que nous attendons toujours. Je le regrette d'autant plus que le projet de loi déposé par votre prédécesseur, M. Franck Riester, madame la ministre, que les députés avaient examiné en première lecture en mars 2020, constituait une solide base de départ. Alors que le Sénat propose, depuis 2015, de rationaliser l'organisation et la gouvernance de l'audiovisuel public en rassemblant ses moyens pour être plus fort sur le numérique, il est paradoxal de constater que c'est le secteur privé qui aura finalement suivi cette voie, avec le projet de fusion entre TF1 et M6-RTL et l'annonce du rapprochement entre Vivendi et Lagardère.

nous avons réussi à le faire évoluer pour en faire une étape utile, en attendant des changements plus ambitieux. Parmi les points qui ont fait l'objet d'un accord avec nos collègues députés, citons les dispositions permettant de lutter contre le piratage.

nous avons dû abandonner en cours de route le mécanisme de transaction pénale, qui faisait pourtant l'unanimité dans la profession. le voeu que ce renoncement de l'Assemblée nationale ne vienne pas affaiblir, dès sa création, le nouveau régulateur, qui aurait ainsi disposé d'un outil efficace et moderne. Au rang des satisfactions, je note que notre commission s'était fortement mobilisée contre le piratage des retransmissions sportives, un sujet sur lequel l'article 3

Je salue la convergence obtenue sur la composition du collège de l'Arcom à l'article 5, qui permet de préserver l'influence du Parlement, à laquelle nous sommes attachés, tout en intégrant la présence de deux magistrats, conformément à la volonté Je vous rappelle, par ailleurs, que le projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution a également fait l'objet d'un accord en La disposition qu'il porte constitue une mesure de coordination nécessaire pour tenir compte du remplacement du Conseil À l'article 10 A, je note l'ajout d'une disposition visant à tenir compte des coûts d'investissement des chaînes historiques lors des renouvellements des autorisations d'émettre. Deux autres avancées concernaient plus particulièrement le service public, l'une relative à la réception du signal local de France 3, à l'article 10 , l'autre à la possibilité d'obtenir des données

après de nombreux échanges, nous avons trouvé une rédaction commune pour l'article 17 , relatif à la réglementation de la production,

Un accord a par ailleurs été trouvé concernant le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales, porté à 19 millions d'habitants à l'article 10 La recherche d'un accord nécessite souvent des sacrifices et nous avons plusieurs déceptions à déplorer. Si nous avons pu intégrer dans le texte l'expérimentation de l'ultra haute définition, ou UHD, nous regrettons l'absence de progrès concernant l'interactivité et la norme, Concernant l'évolution du secteur, nous aurions aimé revenir, à l'article 13 , sur la disposition adoptée en 2016, qui pénalise les opérations industrielles au même titre que les opérations spéculatives. Nous regrettons également Nous regrettons également la rédaction de l'article 13, lequel, à notre sens, comporte un risque juridique en raison d'une disproportion manifeste entre la sanction encourue et les faits reprochés. Avant de conclure, je voudrais en quelques mots replacer notre débat de ce jour dans le contexte plus large de la réforme des relations entre grands acteurs de l'audiovisuel. La transposition par ordonnances de la directive SMA, que nous avons acceptée face à l'urgence, se heurte aujourd'hui, pour être pleinement applicable, à la question toujours épineuse et jamais résolue de la chronologie des médias. Les positions des uns et des autres sont connues il faut maintenant trancher, et chacun doit accepter de faire un pas, pour créer, enfin, le cadre cohérent permettant de poursuivre le financement des oeuvres françaises et européennes.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, cher Laurent Lafon, monsieur le rapporteur, cher Jean-Raymond Hugonet, mesdames, messieurs les sénateurs, les secteurs audiovisuel et cinématographique connaissent des mutations profondes, chacun d'entre nous peut en faire le constat chaque jour. Nos usages changent, avec la multiplication des canaux de diffusion des oeuvres et la possibilité de consommer des offres culturelles à tout moment, sur tout support et en tout lieu. Notre paysage change également, avec l'apparition de nouveaux acteurs géants, aux capacités d'investissement considérables et à l'offre de programmes globalisée, installés en dehors de notre territoire et de sa régulation. Si ces mutations comportent des chances pour la création française, elles appellent aussi à établir de nouvelles règles, adaptées à une économie beaucoup plus ouverte et compétitive. Elles exigent également de trouver les moyens de renforcer notre création et de maintenir une ambition industrielle et culturelle pour et par l'audiovisuel et le cinéma.

J'ai également souhaité que soit déposé le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique. Ce texte important vise à améliorer la protection des droits des auteurs, des artistes, des producteurs, des diffuseurs ou des fédérations sportives, en renforçant la lutte contre le piratage.

d'autant que, après une baisse du nombre de pirates pendant deux années consécutives, les périodes de confinement ont tout récemment favorisé une poussée de la consommation illicite- C'est tout l'objet des premiers articles du projet de loi, qui permettent de dresser une liste noire des sites internet dont le modèle économique repose sur le piratage, de façon à tarir leurs sources de revenus. Ces articles visent aussi à lutter plus efficacement contre les sites miroirs, qui reprennent en totalité ou de manière substantielle les contenus d'un site jugé illicite. Ils créent, par ailleurs, un mécanisme de référé pour lutter contre le piratage sportif. Ce texte permet également la modernisation de notre régulation. La fusion du CSA et de la Hadopi était attendue ; l'Arcom sera dans quelques mois un nouveau régulateur compétent pour l'ensemble du champ de la régulation des contenus audiovisuels et numériques, qu'il s'agisse de lutter contre le piratage, de protéger les mineurs ou de défendre les publics contre la désinformation et la haine en ligne. Ce texte permet, enfin, de garantir l'accès du public à nos oeuvres françaises, en instaurant un dispositif protecteur, qui permettra, en cas de cession d'une oeuvre française, de vérifier que l'acheteur, même s'il ne s'agit pas d'un producteur établi en France, présente toutes les garanties nécessaires pour que l'oeuvre puisse être exploitée et donc vue par le public, en France et à l'étranger.

à l'esprit les dispositions relatives à la modernisation de la TNT, à la redéfinition de la production indépendante, ou encore à l'actualisation des règles anti-concentration pour les télévisions locales et les radios.

L'examen de ce texte s'est déroulé dans un climat apaisé, avec des débats particulièrement intéressants ; ils ont permis qu'un travail de qualité soit mené par vos deux chambres pour l'enrichir. Je veux, à ce titre, chaleureusement remercier le président Laurent Lafon et le rapporteur Jean-Raymond Hugonet de la relation de confiance que nous avons nouée, ainsi qu'avec nos équipes respectives, au cours de cet examen. c'est tout à fait mon état d'esprit : travailler avec chacune et chacun d'entre vous pour faire avancer des chantiers importants pour le secteur de la culture, au-delà des habituels clivages partisans. Grâce à vous, ce projet de loi permettra d'adapter, une nouvelle fois, la loi du 30 septembre 1986 loi du 30 septembre 1986 aux nouvelles réalités économiques et aux nouveaux enjeux de régulation. Il permettra d'apporter des réponses concrètes à trois enjeux essentiels : la protection des droits des auteurs, la modernisation de notre régulation et la défense de l'accès du public aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises,

phase plus tendue de la vie politique, il est utile de rappeler qu'un travail parlementaire peut aboutir, sur des sujets comme la la lutte contre le piratage en matière audiovisuelle. Je me satisfais des avancées que nous avons obtenues et de l'équilibre ainsi trouvé, et notre groupe soutiendra le texte issu de la commission mixte paritaire. La parole

l'ère du numérique a profondément remanié le secteur audiovisuel, en transformant le paysage de la communication, avec ses avancées et ses dangers. Cette mutation est toujours à l'oeuvre, et nous devons répondre aux grands défis qu'elle impose, à savoir la nécessité de protéger les droits de la création,

Il faut en effet agir sur plusieurs fronts, qui sont ouverts tant par la multiplication des types de supports que par la forte croissance des usages, qui ne sont pas tous bienveillants, À cet égard, nous pouvons nous féliciter que le Sénat et l'Assemblée nationale se soient largement accordés sur les dispositifs de lutte contre le piratage, un volet essentiel, puisqu'il touche aux droits de la propriété intellectuelle.

Dans cet esprit, le nouvel article 8 A introduit par nos collègues députés permettra à l'Arcom de contribuer à renforcer la position de la France en matière de protection des droits de propriété intellectuelle auprès des organisations internationales et communautaires.

En première lecture, ma collègue Véronique Guillotin avait rappelé que le groupe RDSE approuvait cette fusion, ainsi que l'élargissement des missions et des pouvoirs d'enquête de l'Arcom. La nouvelle autorité de régulation doit gagner en efficacité pour la protection de la création culturelle et des droits qui en découlent.

En revanche, l'accord trouvé sur le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales et la rédaction renforçant les modalités du nous satisfont. Mes chers collègues, il était urgent d'adapter la grande loi du 30 septembre 1986 aux nouveaux enjeux de régulation d'un paysage audiovisuel renouvelé et fortement traversé par le numérique. Aussi, nous voterons en faveur des textes élaborés par la commission mixte paritaire, lesquels

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme du débat sur ce texte. débat sur ce texte. D'une grande réforme de l'audiovisuel public, nous sommes passés à la protection et à l'accès aux oeuvres à l'heure du numérique, avec comme point central la création de l'Arcom. La télévision traditionnelle voit chaque jour de nouveaux concurrents débarquer pour capter l'attention et les revenus publicitaires qui l'accompagnent. Il est donc nécessaire d'agir, et ce texte porte des avancées, comme toutes les mesures assurant l'effectivité des droits d'auteur et des droits voisins. Nous avons ainsi à l'esprit l'obligation, faite aux fournisseurs d'accès, de prévoir la diffusion des antennes locales sur des numéros de chaînes que je qualifierais de « logiques ». Il n'est pas anecdotique, nous semble-t-il, de donner de la visibilité à nos territoires. nous félicitons également de l'intégration dans les conventions de diffusion de la diversité des pratiques sportives. Nous sommes satisfaits que la CMP ait retoqué l'amende forfaitaire pénale pour piratage, qui risquait, en définitive, de créer un droit au piratage totalement inefficace.

Nous sommes plus mesurés sur la protection des productions. La France ne disposait d'aucun outil de protection des productions françaises, mais la mesure proposée, conçue sous le seul prisme du piratage et omettant le droit des créateurs, répondra-t-elle aux enjeux ? Cela ne nous semble pas

par les pouvoirs publics. S'agissant du piratage, notre groupe rejoint partiellement l'analyse du rapporteur : on doit bien distinguer les piratages individuels des processus industrialisés. L'exemple des diffusions sportives est emblématique. En l'espace d'une quinzaine d'années, la très grande majorité des contenus sportifs, auparavant diffusés en clair, est devenue payante. Cela a conduit non seulement au développement du piratage, mais aussi à un rabougrissement des disciplines retransmises. Or le texte renforce la lutte contre le piratage,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'issue du parcours législatif du présent texte, je ne m'étendrai pas sur la déception qu'a représentée son recentrage post-covid. Chacun l'a souligné, nous attendions une grande loi audiovisuelle, qui avait été annoncée et dont le secteur a aujourd'hui tant besoin, face à un monde qui a changé et qui continue de changer vite, très vite, tout comme le paysage audiovisuel qui se recompose- le rapporteur en a fait état. Le texte qui nous a été finalement soumis n'a pas cette ambition, mais cette version restreinte reste utile, afin de réformer la régulation et la protection de l'accès aux oeuvres culturelles. On notera par ailleurs qu'il a été substantiellement enrichi sous l'impulsion du Sénat. J'en profite pour pour féliciter une fois encore notre rapporteur, Jean-Raymond Hugonet. À l'issue de la commission mixte paritaire, nous nous réjouissons de constater que nombre des apports sénatoriaux ont été conservés,

De même, la détermination d'un compromis concernant le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales va dans le bon sens. Je me réjouis par ailleurs du maintien du principe de modernisation terrestre, qui va permettre, au bénéfice de nos concitoyens, de lancer des services en ultra haute définition et d'instaurer de nouvelles obligations en matière de compatibilité des récepteurs de télévision mis en vente sur le marché. Certains des articles insérés dans le texte par notre assemblée n'ont pas été conservés, mais ont pourtant déjà atteint leur objectif. Tel est le cas de l'article 2 A, qui prévoyait la création d'un régime de gestion collective pour l'exploitation des droits des auteurs d'oeuvres graphiques, plastiques et photographiques. Son insertion en première lecture a accéléré la signature d'un accord entre les artistes graphiques et Google. C'est bien sûr une bonne chose. Je regrette malgré tout la suppression de l'article, car si les contrats ou les accords valent ce qu'ils valent, rien ne vaut la loi gravée dans le marbre. pour l'article 17 , qui prévoyait le maintien de France 4. Après plusieurs années de mobilisation des parlementaires, notamment ici au Sénat, nous avons été entendus Enfin, la possibilité pour l'Arcom de tenir compte des investissements des chaînes lors du renouvellement des autorisations d'émettre entre dans cette catégorie, puisque tel était en substance le sens de l'article 10 , qui a été finalement supprimé. Ces avancées sont notables, mais elles n'interdisent pas d'exprimer des insatisfactions.

Hbb TV, un standard d'interactivité et de diffusion de contenu à la demande, grâce auquel les éditeurs nationaux pourront proposer simplement et directement à leurs téléspectateurs leurs services interactifs. Cette avancée était censée rééquilibrer le rapport de force qui se joue sur la télévision connectée entre les chaînes de télévision et les plateformes vidéo, telles que Netflix, Disney+ et Amazon Prime, dans la mesure où ces dernières disposent des ressources leur permettant de nouer des accords avec les opérateurs et les constructeurs de télévision, pour intégrer leurs applications sur les écrans d'accueil et les télécommandes. Sur ce point important, je déplore que les députés aient décidé de faire marche arrière, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, car cette situation constitue une pratique anticoncurrentielle et nuit à la souveraineté culturelle hexagonale, objectif pourtant affiché du texte. Cette norme est largement répandue dans l'Union européenne. Elle ne pose donc pas de problème au regard du droit européen, comme on veut nous le faire croire. La pression vient des opérateurs, car ils souhaitent continuer à vendre des box. des box. Le coût de cette mise aux normes pourrait être mis à la charge des fabricants de téléviseurs. Contrairement aux arguments que l'on nous a fait valoir, la création à l'article 10 A d'un label dédié à la TNT de nouvelle génération n'est pas une obligation,

ou directive SMA, a marqué une étape majeure dans la modernisation du financement de la création française et européenne, dans un contexte de mutation profonde du secteur audiovisuel.

avancées, qui ont été saluées par les auteurs. Il reste encore des marges d'amélioration. Heureusement, le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas suivi le Sénat sur la dérégulation complète des rapports entre éditeurs et producteurs.

Nous avons fait le deuil d'une réforme de l'audiovisuel public digne de ce nom et saluons les efforts réalisés pour sauver les mesures rassemblées dans ce projet de loi au périmètre resserré. Trois sujets majeurs ont nourri les débats : la création d'une nouvelle autorité de régulation, la lutte contre le piratage audiovisuel et l'accès à l'information et à la culture. Cette nouvelle autorité, l'Arcom, sera dotée de compétences renforcées, avec la création d'une liste noire des sites qui ne respectent pas le droit d'auteur et la possibilité de demander le blocage et le déréférencement des sites miroirs. En matière de piratage, des ordonnances dynamiques d'urgence contribueront à limiter la diffusion de la retransmission illégale de rencontres sportives. Près de 20 % des Français ont recouru au piratage sportif en 2019, notamment des liens diffusés sur les réseaux sociaux. Or les droits télévisés représentent une source essentielle de revenus dans l'économie du sport. Nous aurions pu aller plus loin en matière de lutte contre le piratage de contenus culturels. Le Sénat a proposé l'instauration d'une transaction pénale d'un montant de 350 euros en cas de téléchargement illicite, pour parachever les moyens de lutte contre le piratage. La commission mixte paritaire n'a pas retenu cette proposition, et nous le regrettons. De nombreuses organisations professionnelles sont favorables au renforcement de la réponse graduée et rappellent que le respect du droit d'auteur, sans complaisance, est intimement lié à la liberté de création. Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, j'avais attiré l'attention du Gouvernement sur la persistance de pratiques frauduleuses sur les plateformes musicales. Les manipulations d'écoutes faussent les rémunérations et la visibilité des oeuvres sur internet. Ces pratiques relèvent de l'escroquerie, et il me semble que l'Arcom devrait se saisir de ce problème. D'autres sujets importants ont été évoqués, notamment l'accès à la culture et à l'information. L'une des mesures phares du projet de loi prévoit la création d'un catalogue d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises cédées à un acteur étranger, mais devant rester accessibles au public français. Si le Conseil d'État s'est opposé à la mise en place d'une demande préalable avant toute cession de ces oeuvres, la déclaration préalable permettra à l'État de suivre le respect de l'accessibilité du patrimoine cinématographique français. Enfin, nous saluons la décision du Gouvernement de prolonger la diffusion de France 4. La qualité des programmes éducatifs et culturels de la chaîne permettra, je l'espère, de maintenir sa présence sur la TNT à long terme. Par conséquent, nous voterons ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mais que se passe-t-il dans notre paysage médiatique ?

Dans les rédactions, les plans sociaux se succèdent et les journalistes sont remplacés par des éditorialistes. Dorénavant, les journaux, radios et chaînes de télévision passent de main en main d'un milliardaire à un autre. En achetant des médias, les grands industriels s'achètent de l'influence au détriment de la qualité de l'information et de la démocratie. La concentration des pouvoirs, des opinions et des idées entre les mains de quelques-uns est un glissement dangereux qui s'accentue chaque jour. J'insiste sur ce problème : il est éloigné du texte que nous discutons aujourd'hui, mais, justement, cette loi aurait pu et dû y répondre. Notre corpus législatif concernant le financement des médias date de 1944. La dernière grande loi remonte à 1986. Pourtant, dans ce texte, il n'y a rien qui enraye le glissement en cours dans notre paysage médiatique. Nous avons réussi à maintenir France 4 et Culturebox, ce qui est une bonne nouvelle pour la culture et la jeunesse. Mais sinon, rien ! L'article 10 va même permettre aux chaînes d'information en continu d'ouvrir des antennes dites « locales avec un seuil à 19 millions de personnes, celles-ci pourront couvrir plus d'un quart de la France. Dans les autres volets de ce texte, on manque aussi la cible. On se concentre sur des ajustements techniques, en laissant de côté les questions de fond. Bien sûr, la fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l'Arcom a du sens. Mais cette agence aura-t-elle les moyens d'assurer des missions plus nombreuses et plus complexes ? Sera-t-elle plus efficace que l'actuel CSA pour garantir le pluralisme et le respect de la loi ? Le renforcement du blocage des sites pirates est une bonne chose, mais il est illusoire de penser que cela mettra fin au téléchargement et au illégal. Il y aura toujours des moyens de contournement. Il faut une réflexion globale sur l'accès aux oeuvres audiovisuelles et aux compétitions sportives. L'amende transactionnelle pour les internautes qui téléchargent illégalement a été retirée du texte. C'est heureux, car elle aurait été injuste et inégalitaire. nous allons continuer de dépenser des millions d'euros pour les fameuses « lettres Hadopi », qui sont peu efficaces. Est-ce vraiment une bonne gestion de l'argent public ? Être contre la Hadopi, cela ne veut pas dire défendre le téléchargement illégal C'est simplement reconnaître que cette loi ne fonctionne pas, car elle est facile à contourner. La Hadopi était déjà dépassée il y a dix ans ; elle l'est encore plus aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas convaincue par la rédaction retenue à l'article 17 : les producteurs devront notifier leurs ventes de catalogue au ministère de la culture six mois à l'avance. Il me semble, comme l'avait souligné notre collègue Laure Darcos, que ce délai est irréaliste par rapport aux pratiques du secteur. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'abstiendra donc une nouvelle fois sur ce texte. Notre assemblée doit porter des propositions dignes de ce nom pour répondre à la concentration des médias, car il y a urgence. je vous remercie

nous allons aboutir enfin à l'adoption d'un texte sur l'audiovisuel, après un retard et une réécriture liés en partie à la crise sanitaire, mais en partie seulement, car les hésitations du Gouvernement n'ont pas permis de réaliser la réforme d'ampleur annoncée en début de mandature. Comme je le disais à cette tribune le 20 mai dernier, à l'occasion de l'ouverture de nos travaux, plusieurs big-bangs annoncés à grand renfort de communication ministérielle ont abouti, ces dernières années, à des demi-réformes qui sonnent comme autant de renoncements. Sur ce texte, la déception est d'autant plus grande que l'attente était forte. Je souhaitais ouvrir mon intervention sur cette note négative, car il s'agit d'une occasion manquée sous ce quinquennat de desserrer véritablement le cadre normatif qui contraint le secteur de l'audiovisuel face à la puissance d'action des nouveaux acteurs du numérique. Nous avions pourtant les occasions calendaires et les compétences que le bicamérisme apporte pour construire et voter une réforme systémique, ambitieuse et pérenne. Ce texte ne donnera pas, hélas, à notre audiovisuel, les outils nécessaires pour assurer sa sécurité financière et affirmer son identité de service public, lui permettant ainsi de se confronter aux enjeux nouveaux de la société de l'écran. Le projet de loi initial s'inspirait pourtant des recommandations du rapport sénatorial de 2015 commis par nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin, riche de cette ambition structurelle, mais dont le texte resserré a contraint l'élan réformateur. S'il ne permet pas la réforme globale que nous appelions de nos voeux, le texte que nous examinons aujourd'hui comporte cependant des mesures positives pour soutenir la création et la diffusion audiovisuelles. Ayant participé aux travaux de la commission mixte paritaire, le 1 juillet dernier, je me réjouis que celle-ci ait conservé plusieurs marqueurs essentiels introduits par notre rapporteur Jean-Raymond Hugonet, dont je tiens à saluer la finesse du travail, la détermination courtoise et le caractère précieux de l'écoute, appréciée par ses pairs de tous bords. N'en jetez plus ! Concernant le sujet préoccupant du piratage, le Sénat a renforcé l'efficacité des actions en justice et a étendu le champ d'intervention de l'Arcom. Plusieurs améliorations ont été apportées au dispositif de blocage ou de déréférencement des sites miroirs, ainsi qu'aux mécanismes permettant de lutter contre les sites de sportif. Il est cependant regrettable que l'Assemblée nationale ne nous ait pas suivis sur la voie d'une plus grande responsabilisation des internautes, en refusant qu'une transaction pénale vienne compléter l'actuel mécanisme de riposte graduée. Les chiffres dont nous disposons sont pourtant le signe d'une véritable impunité : en 2020, la Hadopi dénombrait douze millions d'internautes piratant chaque mois, pour un manque à gagner évalué à plus d'un milliard d'euros. Nous veillerons à ce que l'Arcom, nouvelle autorité de régulation aux pouvoirs de contrôle et d'enquête étendus, bénéficie de moyens à la hauteur des ambitions du projet de loi. La création de l'Arcom posait par ailleurs la question de la composition de son collège. Je me réjouis que, en commission mixte paritaire, le Sénat ait pu préserver l'influence du Parlement dans le processus de désignation de ses membres, tout en intégrant la présence de magistrats. Je ne citerai pas l'ensemble des dispositions sénatoriales retenues en commission mixte paritaire, mais je voudrais évoquer les marqueurs me semblant les plus importants. Nous avons permis une meilleure accessibilité de l'offre de proximité de France 3, car il est pour nous fondamental que la télévision publique reflète et accompagne la vitalité de nos territoires. C'est aussi au Sénat que nous devons le maintien de France 4, qui a su démontrer lors du confinement qu'une chaîne de la TNT pouvait porter des programmes de qualité, non seulement divertissants, mais également éducatifs. Rappelons que, avec la suppression de France 4, ce sont plus de 20 % des foyers n'ayant pas accès à l'internet haut débit, qui auraient été privés de ce type de programmes. Nous avons aussi, mes chers collègues, souhaité introduire dans le texte le sujet sensible de la production, afin de rétablir l'équité entre les chaînes historiques et les plateformes numériques. Le compromis trouvé avec les députés doit permettre de réaliser les assouplissements nécessaires en préservant le rôle de la négociation professionnelle. Notre chambre a par ailleurs adopté des dispositions relatives aux autorisations d'émettre des chaînes hertziennes et aux concentrations, afin de permettre le développement du secteur. Concernant le renouvellement des autorisations d'émission, nous avons pu négocier avec les députés la prise en compte par l'Arcom des coûts d'investissement des chaînes historiques, que nous nous devions de soutenir. C'est donc un texte nettement plus ambitieux qui est soumis aujourd'hui à notre vote. Certes, certaines résistances des députés ont conduit à conserver des dispositions nous semblant injustifiées. Je pense notamment à la sanction disproportionnée frappant tout manquement des éditeurs à leur obligation de financement de la production, ou encore à l'absence d'assouplissement du dispositif de lutte contre la spéculation, qui a été adopté en 2016 et qui revient à pénaliser toute opération industrielle. La procédure accélérée ne permettra malheureusement pas de développer de nouveau nos arguments. Par ailleurs, si nous avons pu inclure dans le projet de loi le sujet de l'ultra haute définition, nous regrettons que n'ait pas été maintenu le dispositif adopté par le Sénat visant à développer la norme Hbb TV. Il reste que ce texte est très attendu par les acteurs de la culture et du monde audiovisuel. Il constitue une étape nécessaire, mais non exclusive, pour répondre au défi que représente le maintien de l'exception culturelle française dans un paysage audiovisuel sans cesse renouvelé.

il s'agit d'amendements relatifs à des textes qui ont été promulgués entre les travaux du Sénat et cette dernière lecture,

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

le texte que nous examinons est le produit d'une navette constructive et d'un succès en commission mixte paritaire. Je me félicite du travail effectué par nos deux assemblées. Nous démontrons, une fois de plus, que le climat de coconstruction législative est une garantie d'efficacité de la norme et de sobriété légistique. Notre mission a été de transposer en droit français pas moins de douze directives et quinze règlements européens dans des domaines divers. Afin de traiter la variété des sujets abordés, trois commissions permanentes ont été saisies de ce texte. Aussi, je tiens à remercier mes collègues Hervé Maurey et François Bonneau du travail qu'ils ont effectué, respectivement au nom de la commission des finances et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Bien entendu, il fallait garantir l'exemplarité de la France sur la scène européenne en vue de la présidence du Conseil de l'Union européenne. J'observe qu'il est désormais bien loin le temps où les rapports du Sénat montraient que notre faible taux de transposition, jusqu'en 2000, s'expliquait par une méthode trop technocratique. Aujourd'hui, la concertation en amont et les auditions permettent de mieux prendre en compte l'impact de la norme européenne sur le terrain. J'ajoute que, sous une apparente complexité technique qui a pu rebuter les médias, les implications de ce texte sont considérables, en particulier pour les acteurs des transports et de l'environnement, ainsi que pour nos concitoyens. un seul exemple : quand on plafonne la teneur maximum en soufre des combustibles marins à 0,5 %, on décide, en réalité, qu'un cargo ne pourra plus polluer autant que les 38 millions de voitures du parc français. L'examen de ce texte au Sénat a porté deux ambitions. Tout d'abord, aider les acteurs du secteur des transports à faire face au contexte de crise sanitaire et économique, aggravé par le Brexit. Ensuite, mieux prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement. En première lecture, le Sénat a enrichi le texte de nombreux apports, qui ont été conservés par l'Assemblée nationale. Je pense, par exemple, à la garantie de la confidentialité des tests d'alcoolémie et de substances psychoactives dont pourrait faire l'objet le personnel naviguant à bord d'aéronefs, au renforcement de la lutte contre les « scrubbers », qui génèrent une importante pollution marine au soufre, ou encore aux ajouts opérés à l'article 20, afin de protéger les jeunes marins effectuant des stages à bord des navires, tout en prenant mieux en compte les contraintes du secteur maritime. Plusieurs amendements dits « rédactionnels » ont également amélioré l'intelligibilité de la loi, en supprimant, à la source, des redondances, des articles et des renvois souvent dictés par une volonté de perfectionnisme des administrations d'État. On peut gagner en clarté tout en réduisant l'inflation législative. L'Assemblée nationale a également complété certaines dispositions de manière utile. Je me félicite, par exemple, des modifications apportées à l'article 21 par un amendement du Gouvernement visant à faire remonter la prise en compte des périodes d'activité partielle des marins au titre des cotisations vieillesse au mois de janvier 2021, au lieu du mois de mai, tel que le prévoyait le projet de loi initialement déposé. J'avais moi-même souhaité déposer un amendement en ce sens, mais l'article 40 de la Constitution ne me l'a pas permis. Toutefois, je regrette que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin en neutralisant totalement les effets de la crise sanitaire pour les quelques marins qui seront contraints de reporter leur départ à la retraite afin de ne pas être pénalisés financièrement. Les principales divergences se sont exprimées sur la question des pouvoirs de l'Autorité de régulation des transports (ART). Toutefois, il me semble que la CMP nous a permis de parvenir à une solution de compromis satisfaisante. Le principal point de discussion en CMP a porté sur l'article 6, relatif au secteur aéroportuaire. Au Sénat, notre but a été de renforcer la transparence économique et financière. Nous avons donc proposé d'accroître les prérogatives du régulateur, c'est-à-dire de l'Autorité de régulation des transports, surtout en matière de calcul des redevances aéroportuaires. La sensibilité du sujet a conduit le Gouvernement à présenter des amendements de dernière minute à l'Assemblée nationale. L'explication de fond est simple : comme vous le savez, les opérateurs préfèrent garder leur liberté de manoeuvre et l'État a tendance à vouloir conserver son pouvoir de contrôle. Bref, après avoir tracé un jalon sur la régulation aéroportuaire et obtenu quelques avancées, la sagesse nous a conduits à préserver le succès global de la CMP et à tenir compte du bouleversement du secteur aéroportuaire, en pleine phase de décarbonation, donc d'investissement massif. En 2009, la régulation a été conçue pour que le consommateur puisse bénéficier de hausses modérées de tarifs aéroportuaires. Aujourd'hui, le monde aérien a changé, et la priorité est moins la baisse des prix que la décarbonation. À l'article 13, qui concerne les autoroutes, nous nous sommes conformés aux exigences européennes, tout en sécurisant le champ d'intervention du régulateur. Enfin, les pouvoirs d'enquête de l'ART en matière de transmission d'informations sur les déplacements multimodaux se sont vus consolider aux articles 15 et 15 . Introduits à Introduits à l'Assemblée nationale, ils permettront d'étendre les pouvoirs de collecte d'informations de l'ART aux sous-concessions autoroutières. L'Assemblée nationale a poursuivi le travail engagé par le Sénat, en validant, dès la première lecture, la majorité de ses initiatives ; sur les 42 articles que comptait le projet de loi initialement soumis au Parlement, 40 %- soit 17 articles -ont été approuvés sans modification et 42 %- soit 18 articles -n'ont fait l'objet que de précisions techniques. Au total, il me semble que nous sommes parvenus à un texte d'équilibre, qui permettra à la France de se conformer aux exigences européennes avant la présidence du Conseil de l'Union européenne. La

sont non pas des chimères ou des ambitions lointaines, mais des faits et des réalités tangibles. Régulièrement, des dispositions décidées avec nos partenaires européens viennent enrichir notre droit. Elles créent un cadre unifié en Europe et, ce faisant, permettent de protéger et de renforcer nos industries, nos opérateurs et nos citoyens. C'est le sens du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Après que vous l'avez examiné, ce texte a été complété par l'Assemblée nationale, par exemple sur l'encadrement des prix dans le transport fluvial de marchandises, ou encore sur les mesures relatives aux conducteurs de poids lourds dans le contexte du Brexit. Ces mesures vont dans le sens de celles que vous aviez adoptées, et le fait que la conclusion mixte paritaire ait été conclusive illustre bien cette convergence. Ce texte, je le disais, nous protège. Il protège tout d'abord nos professionnels des transports, tels que nos routiers et nos marins. S'agissant de nos routiers, l'an dernier, l'adoption au niveau européen du paquet mobilité pour le secteur routier a été une avancée considérable, sous l'impulsion de la France.

nous les protégeons de la fatigue, en sanctionnant les entreprises qui ne respecteraient pas le droit au retour des conducteurs, dans leur pays d'établissement ou à leur domicile, et nous durcissons les sanctions en cas de non-respect des conditions de repos. Par ailleurs, nous protégeons nos routiers de la concurrence déloyale, en limitant le cabotage systématique par les transporteurs étrangers. Ces derniers devront désormais respecter une période de carence de quatre jours entre deux périodes de cabotage. Ce projet de loi protège en outre nos marins. Il fait évoluer nos exigences de formation et de temps de travail à leur égard et permet de prendre en compte les périodes partielle pour leurs droits de pension. C'est essentiel à la signature d'accords d'activité partielle longue durée dans le secteur maritime. Le Gouvernement avait d'ailleurs déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour adapter ce dispositif post-covid, en concertation avec les acteurs du secteur. Enfin, ce projet de loi protège davantage les personnels navigants des passagers indisciplinés. Ce texte vise également à renforcer la protection de la planète. Nous allons mieux réguler la teneur en soufre dans les combustibles marins ; nous allons repenser nous allons repenser le service européen de télépéage pour fluidifier le trafic, donc moins polluer ; nous allons renforcer le contrôle des produits mis sur le marché, afin qu'ils respectent les normes environnementales fixées au niveau européen. Enfin, ce projet de loi accompagne nos collectivités et le développement de l'activité sur nos territoires. Il permet d'acter plusieurs avancées importantes. Je pense, notamment, à celle qui est relative au financement participatif, vous avez exprimé une demande d'assouplissement. Les règles actuelles permettent déjà le financement participatif de tout projet soutenu par une collectivité territoriale. Mais des dérogations existent et ont pu être précisées. Gouvernement considère que l'accord trouvé en commission mixte paritaire est équilibré, et je crois, monsieur le rapporteur, que vous partagez ce point de vue. Permettez-moi de revenir sur deux débats à forte composante territoriale que nous avons eus, en particulier au Sénat. En concerne tout d'abord les aménagements liés au Brexit et aux abords du tunnel sous la Manche, ce texte nous permet de régulariser une situation exceptionnelle. Néanmoins, il ne s'agit pas, bien sûr, d'étendre de manière pérenne la dérogation existante à la loi du littoral et au code de l'urbanisme. Cela ne grèvera pas la capacité de développement de Calais et de ses infrastructures. Concernant l'encadrement des aéroports et le rôle de l'ART, plusieurs avancées du Sénat ont été conservées, et le rôle de l'ART a été précisé. l'ART a été précisé. Celle-ci se voit notamment confier une compétence de suivi économique des aéroports, ce qui participera, j'en suis convaincu, au bon fonctionnement et à la reprise du secteur aérien après la crise que celui-ci a connu ces derniers mois. Mesdames, messieurs les sénateurs, d'aucuns reprochent à l'Europe d'être trop abstraite et de ne pas réellement changer notre vie de tous les jours. Les professionnels des transports, les élus de collectivités locales et bon nombre d'acteurs, je puis vous le garantir, verront l'impact concret de l'Europe grâce à ce projet de loi. Et ils le verront très rapidement. Il nous faudra prolonger cet élan. Nous en aurons l'occasion avec la présidence française de l'Union européenne, à partir de janvier prochain. Nous ferons alors des propositions fortes pour mettre fin aux zones grises du droit social européen, notamment dans le transport aérien et maritime. Sur le fret ferroviaire, sur les biocarburants, sur la transition de nos parcs automobiles, nous devons penser et agir encore plus intensément en Européens, pour être efficaces. une Europe qui protège et qui renforce : voilà l'Europe que nous voulons. Voilà l'Europe en laquelle nous croyons et que nous nous efforçons de bâtir inlassablement. De cet édifice européen que nous construisons, ce texte est une pierre. La parole

avec les exigences du droit européen, dans la perspective, comme cela a été annoncé par le Gouvernement, de nous montrer exemplaires au 1 janvier 2022. La présidence française du Conseil de l'Union européenne commencera alors dans un contexte très particulier, marqué par le Brexit, la crise sanitaire ou encore l'urgence environnementale. Si ce texte est essentiellement technique, il n'en comporte pas moins des avancées qui méritent d'être soulignées. Sans refaire le débat qui a eu lieu en première lecture, je rappellerai rapidement quelques-unes d'entre elles, notamment en matière de transports. Résultant de l'adoption du paquet mobilité, des améliorations sont à noter sur les conditions de travail des transporteurs routiers, en vue de préserver leur santé grâce à l'interdiction de la rémunération en fonction de la rapidité de la livraison l'encadrement du cabotage, ainsi que l'application de sanctions à l'égard des entreprises qui ne respecteraient par leur droit au repos. En ce qui concerne les marins, je me réjouis que l'Assemblée nationale ait voté la prise en compte des périodes d'activité partielle pour la validation des droits à pension à compter du 1 janvier 2021, au lieu du 1 mai 2021. pense néanmoins que le Gouvernement aurait pu aller plus loin, pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Enfin, l'ouverture aux collectivités territoriales de la possibilité d'obtenir une délégation de l'État pour l'organisation des lignes d'aménagement du territoire en direction d'autres pays membres de l'Union européenne, reprenant les travaux de la mission d'information sénatoriale sur les transports aériens Les contraintes inhérentes aux transpositions de directives n'ont pas empêché le Sénat de faire oeuvre utile par l'adoption de quelques amendements maintenus par la commission mixte paritaire, tels que la confidentialité des tests d'alcoolémie et de substances psychoactive du personnel navigant à bord des aéronefs ou l'assouplissement de conditions d'accès au financement participatif pour les collectivités territoriales, notamment en leur permettant d'y recourir dans le cadre de tout service public. Pour ma part, je regrette que la législation en matière d'évaluation environnementale n'ait pas évolué de manière à garantir le respect de la directive Projets, alors que la France a fait l'objet de deux lettres de mise en demeure adressées par la Commission européenne. deux raisons à cela : d'une part, les projets qui ont une incidence notable sur l'environnement échappent à l'obligation de procéder à une évaluation environnementale, et, d'autre part, l'absence d'autonomie réelle de l'autorité environnementale. Il reste donc quelques mois pour régler le problème, puisque, semble-t-il, nous serons dans les rails de la parfaite transposition des directives européennes. À cette incertitude juridique s'ajoute un mouvement général de régression du droit de l'environnement qui s'inscrit dans la durée et qui participe à l'instabilité des projets. de l'action publique (ASAP), en date du 30 juillet 2021, réduit la compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP), en abaissant les seuils à partir desquels les équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques doivent faire l'objet d'une saisine. Dès lors, la CNDP considère que 45 % des projets seraient affectés. Autre régression, le décret a également réduit le délai dont dispose l'autorité environnementale pour rendre son avis sur les projets dont cette dernière Alors que la feuille de route française pour l'Union européenne devrait comprendre un important volet de mise en oeuvre du, la conformité de notre législation environnementale me semble primordiale. Malgré cette réserve, le groupe RDSE votera en faveur du projet de loi au regard des ajustements consensuels qu'il apporte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui la fin du parcours législatif de ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, dans le secteur des transports, de l'environnement et de la finance. Ce texte comporte aujourd'hui 49 articles, à la portée très aléatoire. Plus d'un tiers d'entre eux a d'ailleurs été adopté de manière conforme par l'Assemblée nationale. Les autres articles ont été modifiés, le plus souvent à la marge, ce qui fait qu'il ne restait aucun point de désaccord en commission mixte paritaire. Nous l'avons déjà dit en première lecture, le seul objectif de ce texte reste de faire de la France la bonne élève des transpositions avant d'endosser la présidence de l'Union. Si nous comprenons cette stratégie, nous espérons que la présidence de la France pourra, sur ces thématiques, aller plus loin que ce qui nous occupe aujourd'hui, notamment dans le secteur des transports, pour lequel il nous semble urgent de revenir sur le dogme de la concurrence libre et non faussée, qui menace nos services publics et les missions des opérateurs publics. Pour en rester au contenu de ce texte, je souhaiterais rappeler un certain nombre de remarques, qui ont déjà été formulées en première lecture, mais qui restent, à nos yeux, d'actualité. Nous regrettons ainsi toujours les habilitations systématiques à légiférer par voie d'ordonnances, qui privent le Parlement de son pouvoir législatif. Notons également le manque de concertation sur ces dispositions, puisque le Conseil d'État lui-même a déploré « que certaines consultations soient réalisées trop tardivement pour être correctement prises en compte, telle celle de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle Sur le fond, les mesures de ce projet de loi sont largement anecdotiques. Pourtant, certaines nous apparaissent toujours problématiques. Il s'agit notamment du travail des jeunes marins, dont la période de repos se voit rabotée à l'article 20. Pour évoquer encore la question maritime dans sa dimension sociale, nous regrettons la non-prise en compte de toute la période effective d'activité partielle dans le calcul du droit à la retraite des marins. Concernant le secteur aérien, nous regrettons le passage d'un régime d'autorisation à un régime déclaratoire pour les activités aériennes. certaines dispositions sécuritaires, fruits d'un certain zèle, nous paraissent en outre motivées par une volonté de pénaliser les actions citoyennes autour de ces plateformes aériennes. Mes chers collègues, ce n'est pas en muselant la parole que vous obtiendrez le consentement des Français aux politiques menées par ce gouvernement, dans le secteur de l'environnement, où la carence de l'État est reconnue, y compris par le Conseil d'État. S'agissant de ces mesures, et plus particulièrement de l'article 10, il est du reste intéressant de souligner qu'il ne s'agit en rien d'une obligation communautaire. Cet article a suscité une émotion légitime parmi les associations de défense de l'environnement directement visées par ces opérations, telles qu'Extinction Rebellion ou Greenpeace, nous étions d'ailleurs les premiers et les seuls à demander la suppression de ces dispositions. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Enfin, dans le secteur routier, les problématiques du détachement et du cabotage sont évoquées, mais les mesures proposées sont trop timides pour répondre aux enjeux du rééquilibrage modal. Elles confirment la concurrence assez déloyale de la route, faute là encore de moyens au sein des directions concernées pour faire respecter une réglementation déjà bien imparfaite. Mes chers collègues, pour l'ensemble de ces raisons, le groupe CRCE confirme son abstention sur ce texte.

le groupe Union Centriste se félicite que la commission mixte paritaire qui s'est réunie pour examiner ce texte volumineux et technique ait été conclusive, aboutissant à un texte d'équilibre. Il était indispensable de transposer certaines mesures de soutien aux acteurs du secteur des transports, durement affectés par la crise sanitaire et le Brexit, et de mieux comprendre les impératifs de protection de l'environnement. Je pense notamment aux dispositions concernant les échanges transfrontaliers d'informations en matière de télépéage dans l'Union européenne, ou encore à l'encadrement du détachement des conducteurs routiers, qui vise à créer les conditions d'une concurrence plus équitable sur le marché des transports routiers. Notre groupe salue ainsi l'expertise complémentaire des trois commissions permanentes saisies de ce projet de loi, qui ont cherché à renforcer les garanties à l'égard des acteurs concernés, à mieux prendre en compte les enjeux liés à la protection de l'environnement

Je constate d'ailleurs que les apports du Sénat ont été largement conservés par nos collègues députés. Rappelons-le, à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne, nous avions un devoir d'exemplarité en ce qui J'aimerais insister sur ce dernier point : qualifiée de « lanterne rouge » en matière de transposition il y a vingt ans, la France est devenue championne d'Europe dans ce domaine. Pour autant, le législateur doit assurément viser le meilleur équilibre entre sous-transposition et surtransposition, notamment en réduisant les habilitations à légiférer par ordonnances. Ces dernières, en dépossédant le Parlement de ses prérogatives, augmentent d'autant les risques de surtransposition. Enfin, j'aimerais exprimer un léger regret. Alors que la pollution de l'air provoque la mort prématurée de 40 000 personnes chaque année et que le Sénat a évalué le d'une telle pollution entre 68 et 97 milliards d'euros par an, je m'interroge sur les lacunes concernant la transposition de la directive de 2016 relative à la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. la France a en effet été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour le non-respect de cette directive, tandis que, en août dernier, le Conseil d'État a condamné l'État à payer 10 millions d'euros pour n'avoir pas pris les mesures suffisantes en vue d'améliorer la qualité de l'air.

d'une union solidaire qui permette de tirer les acquis sociaux vers le haut. L'Union européenne a plutôt bien réagi face à l'ampleur de la crise sanitaire qu'elle a dû affronter. Je pense au gel des règles budgétaires et au plan de relance européen. La relance européenne est sans doute une chance unique de consolider la construction de l'Union, surtout si nous voulons sortir plus forts de la pandémie, transformer nos sociétés, créer de nouvelles possibilités et répondre ainsi aux impératifs environnementaux.

paritaire consacre de véritables avancées. Parmi celles-ci, il faut citer, dans le domaine des transports, l'amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses ou l'harmonisation des systèmes de télépéage, afin notamment de lutter contre la fraude. Dans le domaine de l'environnement, notons que le texte renforce le régime de sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation sur les hydrofluorocarbures, qui sont très néfastes, la meilleure application de la réglementation européenne en matière de contrôle des eaux usées des installations d'assainissement non collectif ou d'information du public en matière d'environnement, la mise en conformité de notre réglementation avec la directive Habitat en matière de protection de certaines espèces animales capturées ou mises à mort accidentellement, comme les dauphins. dans le domaine de la protection sociale, la traduction, qui était très attendue, de la législation sur les minerais de conflit. Sur ce point, la future directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises loi permettra également une meilleure protection des salariés du secteur des transports routiers, grâce à un meilleur encadrement du travail détaché des conducteurs. Néanmoins, ce texte aurait pu aller plus loin, et nous regrettons certains manques. de la protection des salariés du secteur des transports routiers, nous regrettons que notre amendement, qui visait à ce que les partenaires sociaux aient accès aux données relatives au détachement, ait finalement été écarté. On a invoqué des questions de surtransposition, mais faire avancer l'Union européenne, c'est aussi être capable de prendre le meilleur de celle-ci en optant pour une harmonisation sociale par le haut. Construire une Europe plus solidaire et socialement inclusive permettrait une meilleure adhésion des citoyens. Il y a là un enjeu important pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Si nous approuvons également les dispositions permettant de prendre en compte les indemnités perçues en cas d'activité partielle par les marins

Le Gouvernement aurait pu faire un effort sur ce point et décider de prendre une mesure juste en faveur des métiers difficiles. Demeurent aussi quelques points d'ombre sur les pouvoirs du régulateur dans le domaine aérien.

Or certaines de ces dispositions ne sont pas anodines. Si l'ART est compétente pour fixer les principes d'allocation d'actifs, de produits et de charges, elle ne le sera pas pour fixer les modalités d'application de ces principes. En la privant de cette mission complémentaire et indissociable, elle pourra difficilement juger de la pertinence du niveau des redevances qui lui est proposé. Dans le cas d'une structure comme Aéroports de Paris (ADP), cela pourrait aussi se traduire par des rentes de monopole, donc une surrentabilité.

sur la privatisation d'ADP et la crise sanitaire, la relance de cette privatisation ne serait-elle pas sur les rails ? Dans la même perspective, la possibilité offerte à l'ART de collecter régulièrement des données économiques et financières, disposition adoptée par le Sénat sur l'initiative de son rapporteur Cyril Pellevat,

Les échanges entre le Sénat et l'Assemblée nationale montrent l'importance d'un bicamérisme fonctionnel, particulièrement quand les délais d'examen sont restreints et la technicité du texte importante.

L'adaptation de notre droit interne au droit européen est une prérogative importante du Parlement. Elle l'est d'autant plus dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui commencera, faut-il le rappeler, en janvier prochain. Lors de l'examen du texte en première lecture, j'ai évoqué la mise à jour de notre droit national en prévision de cette présidence. Ma vision reste la même, à savoir des priorités claires pour une autonomie et une souveraineté européennes qui permettront à l'Union de gagner en puissance dans le concert mondial et de protéger au mieux les citoyens européens. Ce texte a mis en lumière des pans essentiels du droit, qui doivent nous servir de boussole lors de cette présidence. Je pense bien sûr à l'environnement, mais également au secteur des transports et à l'économie, sujets si précieux pour les prochaines années, afin d'atteindre les objectifs européens. j'ai aussi défendu plusieurs propositions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, ainsi qu'à notre politique commerciale, avec pour ligne de mire la défense de nos intérêts et de nos valeurs.

Le Brexit est souvent pris en exemple, mais il ne s'agit pas du seul événement ayant des incidences sur la vie des Français. Transposer des directives et mettre notre droit en conformité avec les règlements européens

L'actualité nous l'a tristement confirmé : alors que la directive Oiseaux peine à être appliquée en dépit des demandes de l'exécutif européen, Emmanuel Macron tente de réautoriser les cruelles chasses traditionnelles de plus de 110 000 oiseaux sauvages, au mépris du droit, de l'écologie et des

Une bonne partie de ses dispositions est bienvenue. Je pense au renforcement des prérogatives de l'Autorité de régulation des transports, à l'harmonisation des régimes de responsabilité des transporteurs aériens, au temps de conduite et de repos des conducteurs routiers.

de la procédure, tout d'abord, l'étude d'impact a été finalisée très tardivement, dans des délais contraints, ce qui a rendu le travail du Conseil d'État Sur le fond, ensuite, les restrictions concernant le repos obligatoire des jeunes travailleurs des navires constituent une régression. De même, l'allégement des informations fournies par les sociétés d'investissement lorsqu'elles créent de nouveaux instruments financiers

bien que nous saluions le fait que nous légiférions sur un fléau qui suscite pauvreté, violence, catastrophes écologiques, et profite aux mafias, nous regrettons que les mesures proposées soient trop timides. Le texte prévoit en effet un système de limitation des risques qui repose uniquement sur le devoir de diligence des entreprises. C'est insuffisant au vu des secteurs d'activité et de la puissance des entreprises visés.

Cette disposition relève d'un signal politique outrancier plutôt que d'un souci de sécurité. Désormais, un tel délit sera puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende Pourtant, le délit d'entrave à la circulation aérienne existe déjà. Cette mesure est une réponse disproportionnée aux manifestations qui ont eu lieu pour dénoncer les vols intérieurs et la hausse des émissions de gaz à effet de serre. C'est C'est un moyen détourné d'affaiblir l'action des militants écologistes. Cela fait en outre écho à la récente condamnation d'un journaliste, qui a simplement couvert une action de désobéissance civile. Mais où est donc passée la liberté d'information et de manifester ? Monsieur le ministre, prenez le chemin de la transition écologique. Je vous le garantis : c'est le moyen le plus sûr de limiter l'action des militants écologistes, qui vous font si peur.

mais aussi de la gestion de la crise sanitaire, nous rappellent toute l'importance de la construction européenne et de son accélération. Pour toutes ces raisons, ce projet de loi transpose utilement plusieurs directives européennes et met nos normes nationales en adéquation avec un certain nombre de règlements européens dans les domaines des transports- terrestres, maritimes et aériens -, et de l'environnement, mais aussi en matière financière. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur un grand nombre de dispositions. La commission mixte paritaire, dont j'étais membre, et qui s'est réunie il y a huit jours, a été conclusive. C'est une très bonne nouvelle. Cet état d'esprit collectif irriguera, souhaitons-le, notre présidence au premier semestre 2022. Sur ce texte, donc, un consensus s'est dégagé. Le groupe RDPI votera pour cette version de compromis. Aussi, et sans revenir sur tout ce qui a déjà été dit- nous remercions les cinq rapporteurs des deux chambres pour leur travail -, je souhaite mettre en avant une mesure en particulier,

Fruit d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les collectivités territoriales auront désormais accès à l'emprunt obligataire participatif, et cela sous une forme expérimentale pendant trois ans.

La sécurisation juridique de ce nouvel outil répond aussi à une demande de la Cour des comptes, qui souligne de longue date la nécessité structurelle de diversifier un marché financier aujourd'hui très concentré, et à une volonté forte des élus locaux. L'extension du champ des projets éligibles au financement participatif à tous les services publics, ainsi que la possibilité offerte aux personnes morales d'octroyer des prêts aux collectivités dans le cadre d'un projet participatif sont une avancée majeure pour les élus et les citoyens. L'objectif est également de fédérer la population autour de projets locaux d'intérêt général. La parole

ministre, mes chers collègues, nous achevons déjà l'examen de ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances,

de la défense et des forces armées, saisie pour avis, et, enfin, Hervé Maurey au nom de la commission des finances, qui a bénéficié d'une délégation au fond, ont su identifier les principes cardinaux de ce projet de loi. Aggravation des peines concernant l'intrusion sur les pistes, périodes de repos obligatoire pour les jeunes travailleurs du domaine de la pêche, extension des compétences de l'Autorité de régulation des transports (ART), services de financement participatif, toutes ces questions ont trouvé une réponse appropriée, ce dont nous pouvons nous féliciter. S'agissant des peines sanctionnant l'intrusion sur les pistes, un sujet examiné avec soin en première lecture, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait adopté l'article 10, assorti de corrections rédactionnelles, en considérant que le droit national actuel était insuffisamment dissuasif

Rappelons tout d'abord que cet article vise à adapter le droit français à la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail et à la directive 2017/159 du Conseil

et étendre la période de repos obligatoire dont bénéficient ces jeunes travailleurs de minuit à quatre heures du matin, plutôt que cinq heures. La commission a donc bien évidemment souhaité adopter cet article, tout en y ajoutant une précision bienvenue. Un amendement de Cyril Pellevat tendant à introduire un temps de pause pour les jeunes travailleurs à bord des navires, conformément aux exigences de la directive 94/33/CE, nous défendons la valeur du travail, si essentielle dans notre société, mais nous défendons aussi les temps de pause, lesquels avaient été abrogés par erreur en 2010 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Sur ce point, encore une fois, nous avons obtenu gain de cause. S'agissant maintenant des compétences de l'Autorité de régulation des transports, la mesure très probablement la plus analysée et commentée de ce projet de loi,

en raison de la pandémie. Puisque notre commission s'est toujours montrée favorable à la consolidation des pouvoirs du régulateur, elle a adopté l'article 6, tout en proposant, par l'intermédiaire de notre rapporteur, de permettre à l'ART de collecter régulièrement des données économiques et financières auprès des aéroports relevant de son champ de compétence, afin d'exercer efficacement sa mission d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires. Malheureusement, cette précision n'a pas été conservée, et il eût été dommage de sacrifier un accord en commission mixte paritaire pour cette mesure, fût-elle utile à l'ART. même déception s'agissant de l'amendement de notre collègue Didier Mandelli, qui proposait de confier à l'Autorité de régulation des transports la mission de rendre des avis sur les projets de texte réglementaire entrant dans son champ de compétence. Heureusement, la Haute Assemblée a été écoutée pour ce qui concerne la possibilité offerte à l'ART d'effectuer une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence, et une mission d'information de l'ensemble des acteurs du secteur.

Cependant, compte tenu de la qualité du dialogue entre les parlementaires, l'exécutif et le président de l'Autorité de régulation des transports, notre rapporteur a considéré que cette nouvelle mission confiée à l'ART pouvait être envisagée avec sérénité. Il aurait été étonnant de sacrifier un accord en commission mixte paritaire au motif que nous étions opposés à l'attribution d'une nouvelle compétence à une autorité publique indépendante, alors même que son président lui-même y était désormais favorable.

S'agissant des financements obligataires, c'est-à-dire de la possibilité offerte aux collectivités locales d'émettre des obligations pour leurs projets de financement participatif, le Sénat avait ouvert cette option en première lecture. L'Assemblée nationale l'a supprimée. Nous sommes parvenus en commission mixte paritaire à une solution de compromis : la mise en place d'une expérimentation de trois ans. Je tiens à cet égard à remercier notre collègue députée Aude Bono-Vandorme, rapporteure de la commission des finances, pour nos échanges fructueux et constructifs, qui ont permis cette issue. Les collectivités volontaires pourront donc se porter candidates auprès des ministres en charge des collectivités locales et des comptes publics. Les critères de sélection tiendront à la nature du projet, à son montant, à son coût de financement et, le cas échéant, à son impact environnemental.

Je me réjouis donc que nous ayons pu, par ce texte, améliorer l'accès au financement participatif. Celui-ci permet non seulement d'offrir aux élus un nouveau mode de financement, hors secteur bancaire, mais aussi, et c'est important, de fédérer la population autour de projets d'intérêt général portés par les collectivités locales.

texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un sujet crucial crucial pour ce qui fait l'identité de la France : notre agriculture et l'avenir de nos agriculteurs. Car, comme j'ai coutume de le dire, il n'y a pas de nation forte sans agriculture forte ! De la capacité de nos agriculteurs à dégager des revenus dépend notre souveraineté alimentaire. De cette capacité dépend aussi l'avenir de nos territoires ruraux, de nos paysages, de notre mode de vie. Le sujet de la rémunération des agriculteurs est donc capital. Il l'est parce que la moitié de nos agriculteurs partiront à la retraite dans les dix ans à venir et que la relève a besoin d'un signal clair. Comment s'endetter, même avec passion, sans perspectives de revenus ? l'est aussi parce que l'agriculture n'a probablement jamais eu à affronter autant de défis à la fois : gestion de la ressource, changement climatique, réponses aux attentes parfois contradictoires d'acheteurs se comportant tantôt en citoyens, tantôt en simples consommateurs, le tout dans un monde ouvert, où des modèles agricoles concurrents rivalisent et parfois s'opposent.

LME, qui a porté une dérégulation dans la chaîne agroalimentaire et qui, à mes yeux, confondait d'ailleurs politique sociale de pouvoir d'achat et politique économique agricole.

Les dernières négociations commerciales l'ont bien montré, sans régulation des rapports de force, notre souveraineté alimentaire se trouvera affaiblie. Alors, oui, l'État n'a d'autre choix que d'entrer dans les rapports de force, comme, d'ailleurs, nous l'avions fait lors des dernières négociations commerciales.

dans un bel esprit transpartisan. Je sais pouvoir aussi compter sur le Sénat et la sagesse des sénateurs pour dépasser les clivages sur ce sujet d'intérêt national que constitue l'avenir de notre agriculture.

jamais aisé. Mais c'est aussi un gage de confiance. Or, on ne changera pas la nature des relations entre industriels et distributeurs sans introduire de la confiance, sans garantir aux distributeurs qu'ils peuvent payer plus, parce que les industriels paient correctement les agriculteurs. Nous devons passer de la défiance à la confiance, de relations d'opposition à des relations de collaboration. Ensuite, comme pour toutes relations humaines, intervenir dans les rapports de force suppose une certaine mesure.

Comme nous menons ensemble le combat des clauses miroirs, qui commence à produire ses effets à Bruxelles, nous devons mener ensemble celui de l'origine. Le présent texte, j'en suis convaincu, peut nous y aider.

la souveraineté alimentaire de notre pays. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai entamé cette discussion générale en insistant sur l'aspect capital du sujet. Je sais quelle sur l'agriculture dans cet hémicycle. C'est pourquoi je ne doute pas un instant de la qualité des débats qui auront lieu au cours des prochaines heures. Je voudrais clore mon propos en saluant la qualité des travaux menés par Mme la rapporteure et Mme la présidente

Pour relever ces défis, ils travaillent plus de douze heures par jour, sept jours sur sept. Procédure, malgré leurs efforts, leurs revenus n'ont cessé de diminuer au cours des dernières années. Bon nombre « subissent » une précarité, qui les pousse parfois jusqu'à l'acte ultime, comme l'a souligné le récent rapport de nos collègues Françoise Férat et Henri Cabanel. Ce constat n'est pas nouveau. Pour autant, et en dépit des appels répétés du Sénat à traiter les différentes causes de cette situation- alourdissement des charges, concurrence déloyale de produits importés, pertes de compétitivité les initiatives des dernières années ont échoué à inverser durablement la tendance. Le texte de l'Assemblée nationale n'échappe pas à ce constat. Il ne corrige que partiellement les défauts de la loi Égalim 1, sur lesquels nous avions longuement insisté lors de l'examen de celle-ci au Sénat et dans le cadre du comité de suivi présidé par mon collègue Daniel Gremillet.

Le prix sera déterminé en tenant compte d'indicateurs de référence et pourra fluctuer selon une clause de révision automatique. En aval, l'industriel devra afficher la part des matières premières agricoles dans son tarif fournisseur lorsque ces matières représentent plus de 25 % du volume du produit, cette part devenant alors non négociable. Le prix du contrat pourra lui aussi fluctuer selon une clause de révision automatique. de loi ambitionne de renforcer la « construction du prix en marche avant », en sanctuarisant les matières premières agricoles tout au long de la chaîne de valeur. Enfin, en contrepartie de l'effort de transparence demandé aux transformateurs, il est prévu que les produits dont la construction du prix est dévoilée dans les conditions générales de vente bénéficient d'un principe de non-discrimination tarifaire, c'est-à-dire qu'aucune baisse de tarif ne pourra être exigée par la distribution sans proposer en échange des services avérés. Pour vérifier ceux-ci, un dispositif de « ligne à ligne » est instauré, détaillant avec plus de précision qu'aujourd'hui les avantages commerciaux proposés en échange. Cette proposition de loi, attendue, présente aux yeux de la commission quatre faiblesses, auxquelles nous avons tenté de remédier. Premièrement, elle ne touche que 20 % du revenu agricole

En outre, elle ne dit rien sur les charges croissantes et onéreuses qui affectent lourdement le revenu des agriculteurs. Deuxièmement, cela a été souligné, elle propose un schéma d'une grande complexité, conduisant à tendre encore davantage les relations, voire à ouvrir de nouveaux contentieux., elle s'éloigne de l'efficacité opérationnelle qu'elle prétend viser. Troisièmement, elle déséquilibre la négociation commerciale entre industriels et distributeurs, au-delà de la nécessaire transparence du coût des matières premières agricoles. Elle fragilise en effet le maillon des transformateurs et industriels, en les conduisant à dévoiler toutes leurs marges à la grande distribution. elle porte préjudice à la médiation des relations commerciales, laquelle constitue pourtant une démarche amiable, privilégiée par les acteurs. Face à ces constats, la commission des affaires économiques a tout d'abord renforcé, en le simplifiant, le mécanisme de transparence. Rendu plus opérationnel pour les acteurs économiques, concerne désormais toutes les matières premières agricoles et devient de ce fait plus lisible pour le consommateur et plus impactant sur le revenu de l'agriculteur. La commission a également rééquilibré le rapport de force entre acteurs des négociations commerciales, encadré les MDD qui échappaient à toute « construction en marche avant du prix encadré les pénalités logistiques qui pouvaient être des outils de pressions abusives et renforcé le médiateur pour favoriser le règlement amiable des conflits. Dans le détail, nous avons validé les grandes lignes de la contractualisation écrite, tout en permettant aux interprofessions de donner leur avis avant l'exemption éventuelle de telle ou telle filière. Il convient, en effet, de nous assurer que nous n'adoptons pas aujourd'hui une loi qui sera vidée de son contenu dans les prochains mois. Concernant les relations en aval, nous avons simplifié les dispositifs de transparence au choix du transformateur et élargi le périmètre à toutes les matières premières agricoles, assurant ainsi un niveau de transparence et de sanctuarisation de ces matières, désormais soumises à la non-négociabilité des prix. Ainsi, dans le respect des contrats qu'ils ont signés, les fournisseurs de produits alimentaires pourront afficher la part agrégée que représentent l'ensemble des matières premières agricoles, sous forme d'un pourcentage de leur tarif, ou bien choisir de certifier la part de l'évolution tarifaire découlant de la fluctuation du coût des matières premières agricoles.

Quelle que soit l'option choisie par le transformateur, donc, le coût des matières premières agricoles cranté dans le contrat sera ainsi sanctuarisé dans la négociation. L'option qui contraignait le fournisseur à dévoiler au distributeur le détail des prix d'achat de chacune de ses matières premières du produit, était non seulement complexe, mais donnait au distributeur accès à la comptabilité précise de l'industriel. Nous l'avons donc écartée, tout comme le seuil des 25 %, inéquitable et préjudiciable à l'objectif de meilleure rémunération des agriculteurs. Dès lors que le fournisseur est tenu en amont par un contrat écrit, qui contient une clause de révision automatique des prix, et que cette clause est reprise dans le contrat aval avec le distributeur, l'objectif de traçabilité et de transparence de l'ensemble des matières premières agricoles est atteint. Le distributeur, informé de l'évolution de la part agrégée de ces matières par l'industriel, devra la rémunérer à la hauteur demandée. Pour que l'ensemble du secteur alimentaire participe à la recherche d'une rémunération plus juste de l'amont, la commission a adopté un encadrement des produits vendus sous MDD, soit près de 30 % des denrées, jusque-là exemptés d'indicateurs et de clauses automatiques de révision des prix. Nous avons également renforcé les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles, en lui permettant notamment d'être arbitre, si et seulement si les deux parties en conviennent.

l'objectif pour lequel il a été mis en place, à savoir la meilleure rémunération des agriculteurs, et pas uniquement de ceux qui intègrent les MDD ? Quels sont les effets collatéraux, notamment au regard du cagnottage et des baisses de prix sur les légumes et fruits frais ou sur les rayons détergents et cosmétiques ? Bref, y a-t-il des « victimes collatérales » du SRP ?

Chaque assemblée législative ayant ses prérogatives, il nous appartient, au Sénat français, de respecter le droit européen quand nous écrivons la loi, charge à nous de prendre par ailleurs des résolutions ou de nous exprimer sur les évolutions du droit européen que nous jugeons souhaitables. Nous n'avons donc pas conservé la rédaction de l'article 3 , qui créait une nouvelle pratique commerciale trompeuse, explicitement interdite par le droit européen, donc non applicable en France et, dans l'intention, potentiellement préjudiciable aux entreprises qui « fabriquent en France Afin d'apporter des réponses concrètes et rapides aux abus constatés en matière d'étiquetage, la commission privilégie la transcription du règlement européen à l'article 4, précisant que, si l'origine d'un produit alimentaire n'est pas la même que l'origine de son ingrédient principal, le consommateur devra en être informé de façon explicite.

En l'état actuel du droit, c'est une avancée en matière d'information du consommateur et de protection du logo France. Mais il est évident que le Parlement européen devra revenir sur ce dossier pour répondre aux attentes légitimes des consommateurs. Fort de cette traçabilité opérationnelle renforcée, le texte issu du Sénat devrait permettre de redonner cette valeur tant attendue aux matières premières agricoles, et une plus juste rémunération aux agriculteurs.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'agriculture répond au besoin essentiel de se nourrir, mais elle est également une activité fondatrice de la vie humaine en société. C'est pourquoi, pendant longtemps, les autorités publiques ont fait le choix- j'y insiste -de fixer des prix minimaux pour sauvegarder les intérêts des producteurs en période de surabondance ou, au contraire, des prix maximaux pour protéger les consommateurs des effets de la spéculation en période de pénurie. Il y avait alors une reconnaissance de la spécificité de l'agriculture dans notre société. Puis vint la libéralisation de ce secteur, l'agrandissement des parcelles, l'utilisation massive des produits phytosanitaires et tant d'autres choses lors, notre agriculture connaît une crise, devenue structurelle. Comme pour toute libéralisation, on nous avait promis que le marché garantirait un revenu suffisant aux producteurs, sans qu'il soit besoin de soutiens spécifiques ou de mécanismes de stabilisation des marchés. C'est tout le contraire qui s'est produit : une grande partie des agriculteurs et agricultrices ne parvient pas à vivre du fruit de son travail agricole commune, la PAC, donc les décisions des agriculteurs, en fonction des signaux du marché n'a servi que l'industrie agroalimentaire, dans certaines filières très concentrées, et la grande distribution, organisée, il faut le dire, en véritable cartel. Pis, les gains de productivité dus à l'évolution des techniques n'ont bénéficié ni aux producteurs ni aux consommateurs ; seuls les transformateurs et, surtout, la grande distribution en ont tiré profit. Cette crise est donc la traduction de la libéralisation forcenée.

Elle est la résultante d'un aveuglement, ayant fait des filières agricoles des « chaînes de subordination » dans lesquelles l'exploitant agricole n'est souvent plus qu'un « sous-traitant », comme le disait Fernand Braudel.

au revenu des agriculteurs. En quinze ans, rien n'a changé ! Vous essayez d'imposer le principe de la contractualisation à l'amont de la filière, tout en préservant une certaine forme de flexibilité et tout en étant évasifs sur les contraintes de l'aval. Pourtant, cela fait des années que nous mettons en lumière la nécessité d'indicateurs publics et contraignants, d'un suivi rigoureux des prix et des marges de chacun des acteurs de la filière, de l'établissement d'un prix minimum indicatif pour chaque production, mais aussi d'un prix plancher d'achat aux producteurs, qui doit compléter l'encadrement de la contractualisation. le contrat ne permettra pas, à lui seul, de rééquilibrer une relation commerciale, surtout si les prix doivent être fixés de manière indépendante par chaque producteur ou organisation avec son acheteur.

la libéralisation des échanges, la dérégulation des activités commerciales et le refus de reconnaître une exception agricole. Le constat est aujourd'hui implacable : les coûts de production augmentent, mais les prix payés aux producteurs stagnent ou diminuent, et le revenu paysan continue de se dégrader au profit des grands groupes agro-industriels. Malheureusement, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui ne changera pas fondamentalement la donne. Certes, on peut saluer la création d'un comité de règlement des différends commerciaux agricoles et le renforcement de son rôle après le travail effectué en commission, ou encore la sortie du prix des matières premières agricoles du cadre de la négociation tarifaire entre industriels et distributeurs. Toutefois, comme le soulignait notre ancien collègue Jean Bizet dans son rapport sur l'agriculture et le droit de la concurrence, la contractualisation est privée de l'essentiel de ses effets par le primat donné à la préservation de la concurrence, preuve de la méconnaissance de la spécificité de ce secteur. De plus, il faut s'attaquer à la concentration toujours plus importante de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, porter la nécessité d'un système assurantiel public et universel pour protéger les agriculteurs, un encadrement des prix, une protection du foncier agricole, un soutien à l'installation des agriculteurs ; et la liste n'est pas exhaustive. Surtout, il faut renoncer à la multiplication des accords de libre-échange, qui menacent tout autant l'agriculture nationale que l'environnement. Si nous voulons conserver notre agriculture, nous devons nous en donner les moyens, c'est-à-dire rompre avec la logique libérale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous l'avions dit ici même lors du débat sur la première version du projet de loi Égalim, les dispositions envisagées alors ne régleraient en rien la question de la destruction de la valeur qui doit revenir au producteur agricole. Un an après, la commission des affaires économiques de notre chambre démontrait, chiffres à l'appui, que, pis encore, certaines filières, dont celle du gras, étaient placées dans une situation encore plus dégradée depuis l'entrée en vigueur de la loi. Certains de ses effets ont été corrigés depuis lors, mais, fondamentalement, il n'y a eu aucun ruissellement ou retour de valeur de l'aval vers l'amont. C'est un échec total, et un échec qui était annoncé. Aujourd'hui, avec ce nouveau texte retravaillé par le Sénat, le problème reste entier ou presque. Mais ne nous voilons pas la face : le respect que nous devons aux agriculteurs français nous oblige à leur dire la vérité. La vérité, c'est que l'article 1 de ce texte, outre qu'il ne concerne qu'une part trop faible de la production française, même si le Sénat - je salue à cet égard le travail de Mme la rapporteure et de Mme la présidente a inclus les produits sous marque de distributeur, ou MDD, ne permettra pas de répondre à la seule question qui importe : comment faire en sorte que la vente du produit agricole au premier acheteur soit source d'un revenu couvrant significativement les charges de production Malgré l'favorable de nombre de parties prenantes, on s'achemine vers une nouvelle désillusion. Pour un peu, on penserait que l'objectif premier de ce texte est d'enjamber la période électorale qui s'ouvre La France se dote tous les dix à quinze ans d'une loi sur l'économie. La loi LME de 2008 a érigé en principe intangible la libre négociation des prix. Dans ce cadre, et du fait de sa complexité structurelle, la production agricole n'a pu s'adapter autant que les acteurs de l'aval. En bout de chaîne de valeur, la grande distribution est sortie gagnante de ce rapport de force. Monsieur le ministre, comment, sans aller vers un système de prix totalement administrés, peut-on reconnaître systématiquement aux producteurs agricoles la valeur de leur travail et du capital engagé ? Un texte parlementaire sur les objectifs et les principes qui rendraient nos producteurs et notre économie agricole plus forte, plus résiliente et plus souveraine dans le contexte européen et mondial de la transition environnementale est indispensable et urgent. Monsieur le ministre, la valeur échappe à beaucoup trop d'agriculteurs, et l'on constate, année après année, que les importations s'accroissent sensiblement dans de nombreuses filières, que les exportations, hors vins et spiritueux, sont orientées à la baisse, et, finalement, que le résultat du commerce extérieur agricole s'affaisse. Où va-t-on ? Quelle est votre ambition pour la Nation en matière de souveraineté alimentaire et de reconnaissance du producteur agricole français ? Peut-on en rester là, en laissant jouer les mécanismes darwiniens d'une sélection naturelle des agriculteurs, les petits n'ayant comme perspective que de passer la main, à leur corps défendant, aux mieux portants, et ainsi de suite ? Malgré les apports réels du Sénat, les effets d'Égalim 2 ne seront pas à la hauteur des enjeux pour beaucoup trop d'agriculteurs. Aussi, qu'envisagez-vous donc de faire pour soutenir, malgré tout, le revenu agricole ? Monsieur le ministre, le Gouvernement et le Président de la République projettent-ils une LME agricole, adaptée à notre époque et aux nécessités des transitions, protectrice des agriculteurs français et garante de notre souveraineté alimentaire nationale ? On ne peut pas déconnecter le débat que nous avons aujourd'hui sur la rémunération des agriculteurs de celui sur la PAC, dont l'impact sur notre agriculture restera majeur. Le 4 mai dernier, dans cet hémicycle, les sénateurs socialistes lançaient un débat pour connaître vos intentions concernant le plan stratégique national, le PSN, qui est encore en cours de rédaction. Les règles de ce PSN auront un impact fort sur le revenu de nos agriculteurs. À l'époque, nous vous avions fait part de nos inquiétudes concernant l'élevage, les zones intermédiaires, ou encore la juste prise en compte des territoires à handicap naturel. Nous disions la nécessité d'une PAC plus juste, plus verte et plus résiliente, malgré la baisse sensible de son budget à euro constant. Plus que jamais, nous pensons que tous les leviers possibles doivent être actionnés pour apporter une réponse aux agriculteurs dans la durée : LME agricole, PAC, valorisation des externalités positives de l'agriculture, gestion des risques, souveraineté alimentaire. C'est à l'aune de l'efficacité de ces dispositifs, qui contribuent tous au revenu du producteur, que nous pourrons porter une appréciation censée sur le devenir de l'agriculture française. Égalim 2 est un levier parmi d'autres, dont nous anticipons hélas un effet très modeste sur la rémunération du travail et du capital agricole. En tant que groupe, nous avons malgré tout joué le jeu d'une amélioration du texte issu de la commission. J'espère que nos propositions constructives seront entendues. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un tiers des paysans gagne 350 euros par mois. C'est la moitié de l'allocation du droit d'asile et un tiers du RSA Plus grave, la profession est endeuillée par un suicide par jour. Au rythme des dernières décennies, avec 15 000 disparitions d'actifs agricoles par an, dans vingt ans seulement, les champs français seront totalement silencieux. La loi Égalim de 2018 n'a pas enrayé la baisse de leur rémunération, malgré une augmentation constante des prix en supermarché. Dans un tel contexte, comment redonner l'envie à notre jeunesse de reprendre une ferme ou de s'installer ? Depuis plusieurs décennies, l'agriculture familiale, enracinée, protectrice de la terre et du pays, a été sacrifiée au profit des grands groupes industriels. La responsabilité nous incombe donc de protéger ceux qui nous nourrissent. La transparence totale du coût d'achat de la matière agricole par l'industriel sur chaque produit alimentaire doit être rétablie, tout comme ce texte souhaite imposer l'indication du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires. Je soutiens cette nécessité et je voterai ce texte, quel que soit son format, même si j'espère qu'il sera le plus ambitieux possible. Nous devons notamment aller plus loin en interdisant l'usage abusif du drapeau français sur des produits alimentaires et agricoles non nationaux. entends déjà dire, monsieur le ministre, que ce serait « contraire au droit européen en matière d'étiquetage des produits alimentaires ». C'est là que le bât blesse ! Vous n'avez pas changé de priorité : en préférant la construction de l'utopie européiste, vous détruisez la réalité de la paysannerie française. Nous avons beau légiférer aujourd'hui au Sénat, il n'y a qu'une seule politique agricole aujourd'hui, c'est la PAAC, la politique anti-agricole commune, qui perfuse nos paysans, devenus dépendants de leurs bourreaux En vérité, les paysans veulent vivre non pas d'aides publiques, mais d'une juste rémunération pour leur immense et si précieux travail. Nos agriculteurs, nos paysans, soucieux de la qualité de leur production, donc de la qualité de ce que nous mangeons, ne peuvent être mis en concurrence avec des produits issus des méga-élevages néerlandais, allemands ou polonais. agriculture fait le maximum pour être à la pointe des normes environnementales et sanitaires. La concurrence qui lui est imposée est déloyale. Monsieur le ministre, vous avez par ailleurs tout mon soutien contre ce que vous appelez « l'écologie de l'injonction », qui nous enferme dans l'équation erronée et masochiste « agriculteur-pollueur Les paysans vivent de la nature : ils ne sauraient la saccager ! Je tiens à dire combien les perspectives en matière européenne sont contraires à la protection des paysans de France. La dernière étude du centre commun de recherche de la Commission européenne prévoit des conséquences catastrophiques à la mise en oeuvre du Pacte vert européen : diminution de la production, augmentation des prix, baisse des revenus, perte de la souveraineté alimentaire.

N'oubliez jamais, mes chers collègues, qu'il ne saurait y avoir de pays sans paysans et que de l'avenir de la paysannerie française dépend l'avenir de la France.

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à apporter des correctifs à la loi Égalim. En effet, trois ans après sa promulgation, les effets tant espérés se font toujours attendre. L'équilibre souhaité dans les relations commerciales n'est toujours pas rétabli. La déflation s'est poursuivie, avec- 0,4 % en 2019 et- 0,2 % en 2020. La rémunération des agriculteurs stagne pour certaines filières. Le revenu avant impôt par unité de travail a baissé de 2,5 % par rapport à 2019. On est bien loin d'une revalorisation du revenu agricole ! L'enjeu de la rémunération soulève aussi celui de l'attractivité du métier.

La crise nous a rappelé le caractère fondamental de notre souveraineté alimentaire et le rôle crucial joué par l'ensemble des maillons de la chaîne. Dois-je rappeler que la France n'a connu aucune rupture d'approvisionnement, grâce à nos agriculteurs et à notre industrie agroalimentaire, qui se sont engagés sans relâche ? Rémunérer notre agriculture, c'est préserver notre souveraineté alimentaire et garantir notre indépendance. Notre système ne fonctionne pas suffisamment bien aujourd'hui pour que nos agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Nous dressons donc un constat d'échec. Toutefois,

au profit de la grande distribution et au détriment des producteurs et des transformateurs. Des modifications rapides doivent y être apportées. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui comporte des avancées significatives. Je pense notamment au format écrit du contrat de vente. La pluriannualité du contrat et les clauses de révision sont également satisfaisantes et devraient introduire une plus grande visibilité et plus de transparence.

L'automaticité de la clause de révision des prix en fonction de celui des matières premières constitue un véritable outil. Cet instrument devrait participer à réaffirmer un équilibre entre les acteurs de la chaîne. concerne la non-négociabilité des matières premières agricoles, nous devrons veiller à ce qu'elle soit assortie d'une garantie, afin que les industries agroalimentaires et les transformateurs ne soient pas la nouvelle variable d'ajustement.

les produits alimentaires, dans le cadre d'une renégociation en fonction de l'évolution des prix de l'énergie, du transport ou encore des emballages.

Ainsi, il serait possible d'établir une liste de produits et d'ingrédients primaires exemptés, lorsque leur production ne peut être assurée en France ou que des circonstances particulières causent des pénuries.

Ce sont autant d'injonctions contradictoires, qui grèvent la compétitivité de notre agriculture et, donc, le revenu de nos agriculteurs. Nous devons également nous attaquer à ces sujets.

que celles et ceux qui nous nourrissent ne soient pas rémunérés à la hauteur de la valeur de leur travail ? Comment accepter que, trop souvent, le prix qui leur est payé ne couvre pas même leurs coûts de production ? Au-delà de l'injustice et de la détresse humaine que crée cette problématique, qui suffisent en elles-mêmes à dire l'urgence de la situation, c'est toute notre agriculture qui est menacée. Le revenu des agriculteurs conditionne en effet notre souveraineté alimentaire comment espérer assurer le renouvellement des générations dans un métier où l'on peine à gagner sa vie ? Comment espérer, dans des fermes sans aucune marge de manoeuvre financière, mener à bien la nécessaire et urgente transition agroécologique ? La viabilité et la durabilité de notre agriculture sont une question indissociable de la question du revenu. L'alerte sur ce sujet est lancée depuis de nombreuses années. Déjà, dans le cadre des débats sur la loi Égalim, nous avions alerté sur le caractère trop peu contraignant de ce texte, ce qui rendait improbable un rééquilibrage des relations commerciales. Aujourd'hui, le constat de l'inefficacité de cette loi est largement partagé, et nous nous retrouvons pour un débat Égalim 2,

le travail sur les marques des distributeurs a été renforcé en commission ; la non-négocialibilité des prix agricoles semble intéressante, de même que l'expérimentation d'un tunnel de prix ou d'un « rémunérascore Le texte présente néanmoins des reculs, notamment sur l'affichage de l'origine des produits. Certes, le droit européen nous contraint, mais nous devons trouver des moyens de garantir la transparence pour le consommateur. Nous proposerons des amendements pour améliorer le texte sur ces points. Mais tant que les industriels ou les grandes surfaces pourront se tourner vers des produits importés, tant que les marchés ne seront pas régulés, le rapport de force restera en faveur de l'aval, et le problème restera entier.

Il faut se poser la question de mécanismes permettant d'agir sur les volumes et de réguler les prix, pour garantir une rémunération minimum aux agriculteurs. Par ailleurs, il d'agir sur la demande. Si l'on souhaite une agriculture rémunératrice et écologique, il faut s'assurer qu'elle soit accessible à toutes et tous. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un système à deux vitesses, où les personnes les plus démunies sont contraintes de se tourner vers des produits de faible qualité, à bas coût, et trop souvent importés. Cela passe par une meilleure répartition des aides PAC, notamment par une rémunération des services environnementaux rendus par l'agriculture, qui n'est malheureusement pas prévue dans le futur Plan national stratégique. Cela suppose aussi de limiter les marges de la grande distribution sur ces produits. pense à l'enquête de l'UFC-Que choisir sur la surmarge inacceptable pratiquée pour les produits bio dans la grande distribution. Cela passe aussi par un soutien à la demande locale pour des produits de qualité et rémunérés équitablement. C'est pourquoi nous défendons avec force dans les textes budgétaires le renforcement des projets alimentaires territoriaux,

également de mettre en oeuvre rapidement le chèque alimentaire durable, qui devrait à nos yeux constituer la base d'une réflexion pour la création d'une sécurité sociale de l'alimentation garantissant à la fois un droit à une alimentation de qualité et des revenus décents

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est très attendue par le monde agricole, car elle vise à protéger la rémunération de nos agriculteurs. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'ambition affichée par le Président de la République depuis le début du quinquennat : permettre à chacun de vivre de son travail. Or, on le sait bien, le revenu des agriculteurs ne reflète souvent pas les efforts et le travail qu'ils fournissent au quotidien. Aussi, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, c'est avant tout leur garantir l'obtention d'un prix rémunérateur. Tel n'est pas toujours le cas. En effet, dans le cadre des négociations commerciales au cours desquelles se déterminent les prix, nos agriculteurs sont souvent le plus faible des maillons de la chaîne les liant aux industriels et aux distributeurs. Il s'agit donc de rééquilibrer ces relations, de manière à assurer un partage plus équitable de la valeur entre les différents acteurs. La loi Égalim de 2018 avait fourni pour cela des outils efficaces, pour peu qu'ils soient utilisés. Si elle n'a pas permis d'atteindre les résultats espérés, elle a toutefois le mérite d'avoir encouragé les interprofessions à se structurer et se renforcer, tout en esquissant une nouvelle logique d'élaboration du prix. Il nous faut aujourd'hui aller plus loin, tirer les leçons de la loi Égalim et parachever ce qui a été entamé. Pour ce faire, la proposition de loi du député Gregory Besson-Moreau vise à sanctuariser les coûts de production dans l'élaboration du prix de manière à garantir aux agriculteurs un prix rémunérateur. Plus largement, il s'agit d'organiser les relations entre les différents acteurs, de l'amont à l'aval de la chaîne alimentaire, en y introduisant une plus grande transparence, pour plus de confiance entre les acteurs. Nos débats en commission ont fait émerger quelques sujets de crispation. En effet, le texte, tel qu'il est issu de la commission, nous semble remettre en cause l'équilibre fragile auquel était parvenue l'Assemblée nationale. Tout d'abord, concernant la question du seuil, il a la réécriture de l'article 2, à la suppression du seuil de 25 %. Il s'agissait d'indiquer, chaque fois qu'une matière première agricole représente plus de 25 % du volume du produit, sa part dans le tarif du fournisseur. Ce seuil de 25 % permettait de donner la priorité aux produits agricoles

on peut discuter de certains ajustements, mais l'existence de ce seuil nous semble essentielle. C'est ce que nous défendrons lors de nos débats. À l'article 3, les modifications adoptées concernant le comité de règlement des différends commerciaux ont pour effet de substituer au recours à ce dernier la saisine du juge. Cela pose selon nous un problème de lisibilité du droit, qui nécessite une clarification. est par ailleurs revenue sur l'interdiction des pratiques trompeuses en matière d'indication du pays d'origine sur les produits alimentaires. Or cette interdiction est une demande forte des agriculteurs, qui considèrent ces indications comme un gage de qualité et de compétitivité. le dispositif initial peut être amélioré dans le but de ne pas pénaliser nos fabricants, dont certains recourent à des produits agricoles que l'on ne trouve qu'à l'étranger,

RDPI espèrent donc une évolution du texte résolument tournée vers nos agriculteurs. Sans évolution notable à l'issue de la séance, nous choisirons de nous abstenir.

Notre travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Comment être rentable lorsque les prix de nos productions sont les mêmes qu'il y a trente ans, alors que les charges n'ont pas cessé d'augmenter ? La plupart d'entre nous vendent à perte.

Cette proposition de loi offre un débat- un débat de plus ... Ce que les agriculteurs attendent, ce sont des actes et des solutions afin d'atteindre un objectif clair : un véritable partage, décent, de la valeur. était d'ailleurs l'objectif annoncé de la loi Égalim. On l'a vu, on le voit, le compte n'y est pas : je rappelle que 20 % des agriculteurs n'ont aucun revenu. Si j'ai soutenu l'idée de mettre toutes les parties prenantes autour d'une même table et si j'ai, avec d'autres, participé aux États généraux de l'alimentation, car la méthode était bonne, je regrette que celle-ci ait été abandonnée très rapidement.

Les enjeux étaient très bien posés, les objectifs étaient clairs et la méthode était bonne. Qu'a-t-il manqué ? Tout simplement le sens de la réalité ! Dans un marché mondialisé, en effet, les agriculteurs sont des pions. Pièces centrales de la chaîne, sans qui rien ne peut aboutir, ils sont pourtant les plus précaires, car ils dépendent du bon vouloir de leurs partenaires. Aujourd'hui encore, ils ne fixent toujours pas le prix de leur production

les distributeurs et les industriels ont négocié leur propre relation commerciale, l'objectif étant l'attractivité pour le consommateur. La guerre des prix peut commencer avec, dès le départ, un déséquilibre et un lien non sincère qui pipent les dés au seul détriment des agriculteurs.

Personne ne peut réellement comprendre le désarroi de la profession : aux prix non rémunérateurs s'ajoutent régulièrement les catastrophes naturelles. Nous en avons vécu une cette année, la gelée noire. Le paysan a pleuré deux fois

nous continuons à chercher quelle loi pourrait permettre aux agriculteurs de vivre mieux ... Selon moi, il faut de véritables mesures coercitives. En 2008, la loi de modernisation de l'économie (LME) a libéralisé les relations commerciales- vous l'avez rappelé, monsieur le ministre. Elle est à l'origine de la guerre des prix menée par les enseignes de la grande distribution, et ce, chacun le sait, au détriment des agriculteurs. Son impact n'a certainement pas été suffisamment mesuré. C'est la LME qui a permis la concentration des coopératives d'achat et resserré l'étau autour des paysans. Si nous comprenons l'enjeu politique que représente le maintien du pouvoir d'achat du consommateur, il faut aussi poser les enjeux de l'avenir de notre agriculture. Sachant que la moyenne d'âge des agriculteurs est de 55 ans, comment intéresser les jeunes ? Comment leur donner envie de s'installer en l'absence d'une véritable vision partagée ? Cette proposition de loi comporte quelques mesures positives, comme la non-négociation du prix des matières premières. Règlera-t-elle pour autant la problématique de la rémunération des agriculteurs ? Réformons la LME : c'est l'une des solutions. À l'heure où l'e-commerce a su se saisir des perspectives du marché alimentaire, notamment celui du bio, il est urgent d'agir.

Cette situation, dont nous sommes les témoins au quotidien sur nos territoires, doit nous faire réagir et nous inciter à modifier lois et règlements pour aider les agriculteurs. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Les raisons de ce mal-être sont multiples et certaines d'entre elles sont bien identifiées : une pression à la baisse sur les prix, accentuée par le secteur de la grande distribution, qui se répercute sur l'industrie, elle-même exerçant une contrainte sur les conditions de marché accordées aux agriculteurs.

Le déséquilibre des négociations commerciales au détriment des producteurs agricoles place ces derniers en position de « preneurs de prix ». On l'a dit, leur mauvaise rémunération a des conséquences désastreuses sur la santé économique des exploitations, mais aussi sur le moral des agriculteurs.

Ce texte est incontestablement un progrès par rapport à la loi Égalim 1, même si les règlements européens nous empêchent encore d'aller aussi loin que voulu et que nécessaire. La grande distribution capte 75 % des dépenses alimentaires des Français. Malheureusement, certains acteurs du secteur ne participent pas autant qu'attendu à la revalorisation des filières agricoles. Le Gouvernement et le Parlement ont fait des propositions, notamment la commission d'enquête du groupe UDI et indépendants de l'Assemblée nationale ou le travail de Serge Papin, chargé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'un rapport concernant les relations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs. de loi que nous examinons aujourd'hui reprend des dispositifs figurant dans les deux rapports issus de ces travaux. Je pense notamment à la pluriannualité des contrats et aux méthodes de règlement des différends commerciaux est aujourd'hui d'obtenir une plus juste rémunération des agriculteurs, qui exercent un métier difficile et primordial pour notre souveraineté alimentaire. alimentaire. L'article 1, qui a pour but de rendre obligatoires les contrats pluriannuels entre producteur et premier acheteur, constitue une avancée. Il permettra au producteur d'avoir une vision à plus long terme sur sa production.

L'article 2, qui prévoit un affichage destiné au consommateur sur les conditions de rémunération du producteur, est sans nul doute important. les consommateurs ne connaissent pas le prix des matières premières qui composent un produit fini ; or c'est ce prix qui est depuis trop longtemps tiré à la baisse. L'article 3, qui limite l'utilisation du drapeau français et de la mention « Fabriqué en France » afin d'interdire les pratiques commerciales trompeuses, est nécessaire, mais doit être plus précis. Tel est l'objet de la modification apportée par le Sénat.

pas. On s'attaque ici au prix de vente des produits agricoles et aux revenus des agriculteurs ; malheureusement, l'effet attendu de la loi ne concernera que 20 % à 30 % de la production agricole.

les produits français ne sont souvent pas compétitifs. Notre agriculture fonctionne à deux vitesses : l'agriculture qui est sans doute

Les agricultrices et les agriculteurs ne perçoivent toujours pas la juste rémunération qui leur est due. Pourtant, ils sont près de 400 000 à travailler chaque jour pour garantir notre autonomie alimentaire : ils sont près de 400 000 à se consacrer à la production de denrées de qualité qui font la fierté et la réputation de nos territoires. en valeur à près de 76 milliards d'euros, la France reste le premier producteur agricole de l'Union européenne. Un peu plus de 50 % du territoire de l'Hexagone est couvert de surfaces agricoles. L'agriculture est donc à la fois un enjeu économique et un maillon essentiel de notre aménagement du territoire. Mes chers collègues, vous le savez, la situation est grave. Le nombre d'agriculteurs diminue, les exploitations peinent à trouver repreneurs la faute à un système qui ne reconnaît pas le travail, la faute à un système qui continue de privilégier industriels et gros distributeurs, la faute à un système libéral où la concurrence et la guerre des prix font la loi. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens ; son adoption à l'unanimité à l'Assemblée nationale l'atteste. Cependant, est-elle à la hauteur des enjeux, de l'urgence, ou n'est-elle qu'un outil sans lendemain, une fois passée la période électorale ?

par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués restent en deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession. Le dispositif proposé dans cette proposition de Tant que la couverture des coûts de production des agriculteurs ne sera pas garantie dans les négociations commerciales, leurs revenus non plus ne pourront être garantis. Ces négociations devront également prendre en compte la rémunération de la main-d'oeuvre agricole afin d'être au plus près des réalités. C'est ce que nous proposons. Mes chers collègues, nous devons protéger davantage nos agriculteurs. C'est pourquoi le groupe SER propose de plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d'erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle. En effet, les taux de service imposés par les distributeurs sont en moyenne de 98,5 % et peuvent atteindre 99,9 %. Ces situations génèrent automatiquement l'application de pénalités, qui deviennent quasi systématiques et sont insoutenables En outre, parce que la transparence doit être une priorité pour donner davantage confiance aux consommateurs, nous proposons de rétablir l'esprit de l'article 3 , qui a été vidé de sa substance en commission. Il faut réaffirmer la nécessité de s'opposer aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires, afin d'assurer aux consommateurs une information claire et fiable. Mes chers collègues, je l'ai déjà dit, cette proposition de loi va dans le bon sens. Cependant, elle ne suffira pas. La politique des petits pas a assez duré ! Face à l'urgence de la situation, une réforme d'ampleur est nécessaire pour poser pour poser les cadres d'une nouvelle grande loi économique, adaptée à son époque. Nous devons travailler à préserver l'agriculture française ainsi que notre souveraineté alimentaire.

et encore moins sur les charges ! Vous ne parlez pas de la problématique de la main-d'oeuvre en France, qui est 1,5 fois plus chère qu'en Allemagne, 1,7 fois plus chère qu'en Espagne et x fois plus chère que dans les pays de l'Est ! Rien sur les charges, donc ; pourtant, Égalim 1 a créé des charges supplémentaires, qu'on a facilement

sécuriser la part agricole dans le tarif du fournisseur et améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs- ce rapport de force est aujourd'hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME.

la mise en place d'indicateurs et d'outils indispensables à la construction de contrats et de prix équilibrés. Toutefois, des difficultés persistent, l'évaluation du coût du produit agricole dans le prix de revient du produit alimentaire. Les mesures prévues ne permettent malheureusement pas d'envisager une réelle maîtrise des charges et dépenses. Par ailleurs, l'ensemble de ces dispositions n'entraîneront-elles pas une augmentation du prix du produit,

ils nous accusent de les abandonner. Comme disait Franklin Roosevelt, « les gagnants trouvent les moyens, les perdants des excuses » ! Égalim 2 ne doit pas être une illusion, un mauvais d'Égalim

l'ambition du législateur était une meilleure redistribution de la valeur. Nous en voulions le ruissellement ; or les producteurs ont vécu un tarissement de leurs ressources. Il convient aujourd'hui de saluer la volonté de corriger les incomplétudes et les insuffisances du texte initial. Rendre obligatoire la contractualisation des accords est indispensable ; mais nous devons accompagner les David de la négociation commerciale confrontés aux Goliath de la grande distribution. Les jeunes agriculteurs nous disent que « le diable se cache dans les détails » et que « les contrats sont des combats nous devons donc légiférer jusqu'à une formalisation précise des clauses constitutives et de leurs révisions. Nous devons imaginer un outil normalisé qui conjuguerait la souplesse de la négociation avec la nécessité de se conformer à une série de composantes auxquelles on ne pourrait déroger. Néanmoins, il serait naïf de croire que le contrat pluriannuel garantirait un engagement tenu. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles doit être doté d'un arsenal de sanctions suffisamment dissuasif, en adéquation avec la nature du préjudice. En effet, la nécessaire médiation ne permet que rarement la résolution des conflits. Je soutiens la nécessité d'imposer la transparence du calcul des prix et d'en garantir une stabilité relative. Je soutiens la volonté de mettre fin à l'obscurantisme de certaines pratiques. Pour autant, ne négligeons pas le rôle majeur du consommateur dans la chaîne de valeur. En effet, la transparence et la non-négociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires doivent se traduire par une lisibilité sur l'étiquetage des produits. L'introduction de 2 % d'huile de lin dans l'alimentation porcine ne fait pas de la charcuterie un produit riche en oméga 3 ! L'affichage d'un drapeau bleu blanc rouge ne certifie pas forcément l'origine française ! La tromperie du consommateur ne doit plus être tolérée Changeons de regard sur le consommateur ordinaire : il n'est pas un perdreau de l'année ... Nous pensons de manière réductrice que l'est la victime inconsciente du marketing. Permettons-lui de prendre des décisions éclairées. Donnons aux Français les moyens de faire des choix et la capacité de réaliser des arbitrages. Les indicateurs de coût de production et de niveau de rémunération doivent contraindre les loups de la grande distribution à entrer dans une dynamique vertueuse et nous permettre de mettre fin au subterfuge des marques de distributeur, les MDD. Affichons les provenances, au-delà de la labélisation France. Informons les consommateurs de l'origine des produits et de la provenance des composants intervenant dans la transformation, sans avoir besoin de démontrer « un lien avéré entre certaines propriétés des produits agricoles et leur origine

Nous estimons que seules une réforme d'ampleur et une remise à plat complète permettront d'inverser les rapports de force dans les relations commerciales, principalement en ce qui concerne

Il n'en reste pas moins que la logique très ou trop libérale ayant guidé la loi LME est encore prépondérante. Par cet amendement, nous vous proposons

pour une réforme d'ampleur posant le cadre d'une nouvelle grande loi économique adaptée à son époque, au regard de la nécessité de préserver l'agriculture française et notre souveraineté alimentaire, tout en prenant en compte les nouvelles contraintes

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue tout d'abord l'opportunité qui nous est donnée de renforcer la loi Égalim pour améliorer le revenu des agriculteurs et rééquilibrer autant que possible les rapports de force entre les fournisseurs et les distributeurs.

la place des transformateurs et des fabricants français est essentielle. Ces petites et moyennes entreprises représentent 98 % des entreprises agroalimentaires. De plus, elles privilégient l'approvisionnement local et les circuits courts, ce qui est un élément majeur pour l'économie nationale et les emplois dans nos territoires. Je me réjouis, à cet égard, que la commission ait adopté ma proposition de simplification concernant la facturation des fournisseurs. Le texte voté à l'Assemblée nationale prévoyait l'obligation de faire apparaître des informations, mais, dans les faits, une telle C'était une demande forte et légitime de ces PME ; je remercie Mme la rapporteure d'y avoir répondu favorablement. Toutefois, une forte inquiétude demeure parmi ces entreprises sur l'impossibilité de répercuter leurs coûts de transformation des produits dans le tarif de vente au distributeur. Dans mon département, plusieurs d'entre elles m'en ont fait part, qu'il s'agisse de boulangers, de torréfacteurs, de charcutiers-traiteurs ou de marques bien connues de chocolats et de confiseries. La crainte est forte de n'être qu'un maillon de la chaîne, sans pouvoir de négociation. Il faut Il faut éviter que ces PME ne soient prises en étau entre, d'un côté, la variation des tarifs des matières premières et, de l'autre, l'impossibilité de répercuter leurs coûts sur les prix de vente. Il est impératif qu'elles restent compétitives. Il s'agit, pour beaucoup, de petites et de moyennes structures, qui ne doivent pas disparaître des linéaires en laissant la place aux multinationales de l'agroalimentaire. C'est pourquoi j'ai souhaité redéposer un amendement à l'article 2 D, dans l'objectif d'intégrer durablement les transformateurs de l'agroalimentaire dans les négociations, comme nous le faisons avec les producteurs agricoles. La parole est à M. Fabien Gay,

lors des négociations d'accords de libre-échange, sur le modèle de l'exception culturelle. Il ne pourra pas y avoir d'équilibre dans les relations commerciales tant que l'agriculture sera banalisée. Il ne pourra pas y avoir de revenu décent pour les travailleurs de la terre ou de révolution écologique tant que nous resterons dans une logique concurrentielle. La nourriture est un besoin humain ; à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. Notre souveraineté alimentaire ne peut en aucun cas constituer une monnaie d'échange. Le XXI siècle présente des défis climatiques et alimentaires que nous avons le devoir et la responsabilité de relever pour préserver notre planète et ses ressources. Or les nouveaux traités bilatéraux, à l'exemple de

dans le Mercosur, tout le bétail est nourri aux OGM et l'utilisation du glyphosate n'est pas réglementée. Un quota d'importation de viande ovine sans droits de douane entraînerait donc des coûts moindres ; nos éleveurs ne pourraient pas rivaliser, sauf à rogner sur la qualité et l'éthique. Il en est de même avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Pourtant, lors des discussions sur le projet de loi Égalim 1, madame la rapporteure, et nous étions d'accord avec vous, vous aviez exprimé votre regret que l'agriculture soit trop souvent une variable d'ajustement. Vous aviez dénoncé le manque de réciprocité des normes de production ; il semble bien que vos inquiétudes et les nôtres soient légitimes. Le ministre d'alors nous avait répondu comme vous, monsieur le ministre : clauses miroirs ! Pourtant, les produits alimentaires importés dans l'Union européenne ne respectent pas toujours les mêmes normes que celles qui sont appliquées dans l'Union européenne.

La crise a aussi montré la nécessité d'assurer notre souveraineté alimentaire, qui est vitale pour notre sécurité sanitaire et environnementale. Nos filières agroalimentaires doivent redevenir une force économique nationale. Pour ce faire, il est indispensable que les agriculteurs français perçoivent le juste prix rémunérateur de leur production. Les agriculteurs attendent des solutions concrètes et pérennes. En 2017, les États généraux de l'alimentation ont créé des espoirs de rémunération plus juste pour les producteurs. Le Sénat l'a souligné, la loi Égalim n'a pas apporté les résultats escomptés. Aujourd'hui, ce nouveau texte est une occasion de renforcer la loi Égalim et de sécuriser la part agricole dans le tarif du fournisseur afin de réellement construire des prix en marche avant. Certaines dispositions sont intéressantes. Il convient notamment d'être particulièrement attentif à la contractualisation, rendue obligatoire et pluriannuelle.

Vous êtes le ministre de l'agriculture. Il faut faire confiance à nos agriculteurs et maintenir la diversité des agricultures sur notre territoire. Donnons à notre agriculture les moyens de tenir et de se développer. C'est l'intérêt de notre pays. Nous serons vigilants sur ce texte

qui l'empêchera d'avoir l'effet escompté. Au vu du déséquilibre actuel des rapports de force dans la chaîne de production agricole, tant que la couverture des coûts de production des agriculteurs ne sera pas garantie dans les négociations commerciales, le revenu de nos agriculteurs ne pourra pas non plus Comme nous l'avons déjà indiqué, si cette proposition de loi prévoit certaines avancées, il n'en reste pas moins que son efficacité en termes de revenus des agriculteurs est loin d'être assurée. À titre d'exemple, ainsi que l'ont rappelé les représentants de certaines structures que nous avons auditionnés, dans le secteur de la viande bovine Label rouge, où la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués sont restés en deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession. La couverture des coûts de production est donc indispensable ; cette position est défendue depuis plusieurs années par le groupe socialiste du Sénat. On nous rétorquera, bien évidemment, que nous ne sommes pas dans une économie administrée ou encore que la couverture des coûts de production pourrait se transformer en prix plancher Nous avons conscience des risques induits par cet amendement. Toutefois, nous estimons que la rédaction actuelle de la proposition de loi comporte de nombreux risques, particulièrement en en termes d'inefficacité sur le revenu des agriculteurs. En conséquence, nous préférons aller de l'avant et proposer des dispositifs plus ambitieux. Les deux amendements

cela doit être pris en compte, non une formule magique imposée par l'industriel lors de la discussion, mais bel et bien par les agriculteurs, leurs représentants, les organisations syndicales et professionnelles.

En ne votant pas cet amendement, nous reconnaîtrions qu'il est possible, au nom de la concurrence, de payer un agriculteur en deçà d'un prix couvrant ses coûts de production.

que les dispositions relatives aux contrats écrits, dont celles qui sont relatives aux modalités de détermination et de révision des prix, ne s'appliquent pas aux coopératives si leurs statuts ou leur règlement intérieur « comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses

Or tous les produits transformés à la ferme ne sont pas forcément vendus directement au consommateur. Certains d'entre eux peuvent intégrer de nouveaux circuits, tels que le e-commerce ou, de façon plus régulière- on le voit de plus en plus -, l'approvisionnement en circuit court de la restauration collective. Cet amendement vise à couvrir un champ plus large des nouvelles pratiques commerciales, en y ajoutant les ventes de produits transformés à la ferme, et permet de « coller » à l'actualité en termes de commercialisation de produits agricoles.

La diversification des productions et des débouchés constitue un enjeu prioritaire de création de valeur pour les agriculteurs. Les circuits courts répondent à une demande des consommateurs quant aux objectifs de politique publique d'approvisionnement en restauration collective et permettent une meilleure maîtrise de son prix par l'agriculteur. De ce fait, au-delà des circuits courts, cette diversification implique d'élargir la terminologie de vente directe La commission a fait remarquer que la rédaction de cette disposition n'était pas encore aboutie. Nous souhaitons néanmoins mettre le sujet en débat, car il paraît important de lever les obstacles au développement des circuits courts,

? Ces amendements identiques visent à élargir les possibilités pour un producteur agricole de déroger aux règles d'apport total de leur organisme de production.Cela

En l'état, il exclut simplement de la contractualisation écrite les produits transformés à la ferme, mais il n'agit pas sur la règle d'apport total et sur la possibilité d'y déroger pour certains produits. produits. Or les produits vendus en circuits courts, s'ils relèvent de la vente directe aux consommateurs, sont déjà exclus de la contractualisation écrite. Compte tenu du caractère réglementaire de ce sujet, j'imagine que le ministre va nous indiquer quelle suite il entend